La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 7 mars 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été publiée.

visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte part d'un constat désolant, mais lucide ; d'un constat qui prend ses racines dans des années où le maintien de l'ordre a changé.

Depuis les sommets internationaux jusqu'aux manifestations du 1 mai, depuis la loi El Khomri jusqu'aux événements les plus récents, la doctrine de maintien de l'ordre est en profonde mutation. à chaque occasion, des brutes s'infiltrent dans les cortèges. Elles pillent les commerces, détruisent le mobilier urbain, attaquent les forces de l'ordre. Elles s'en prennent aux institutions et défient la République. changent les manifestations en émeutes. Ils blessent policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, manifestants. Au fond, ils sont la plus grande menace pour le droit de manifester. C'est bien de cela que nous parlons,

le ministère de l'intérieur a le devoir de protéger le droit à manifester en sécurité. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette question, vous la connaissez bien. Vous l'avez étudiée, comprise. Vous avez choisi de réagir dès juin dernier en offrant de nouveaux outils aux forces de l'ordre, à la justice et aux préfets. Vous avez pris les devants et, avant même les manifestations des « gilets jaunes »- il est important de le préciser -, vous avez proposé d'agir afin que les forces de l'ordre aient toutes les cartes en main pour protéger nos concitoyens. Je tenais donc à saluer l'initiative du président Retailleau. C'est grâce à elle que nous pouvons examiner ce texte et nous donner les moyens d'agir contre les individus violents,

le ministre de l'intérieur, qui veut donner aux préfets et aux forces de sécurité le cadre administratif et juridique adapté pour protéger ; le ministre de la sécurité et des libertés, qui veut rappeler que toutes nos procédures, toutes nos actions, toutes nos décisions sont guidées par deux principes : nécessité et proportionnalité.

de protection pour les manifestants, qui sont pris en otage par les casseurs, par ceux qui cherchent le chaos,- les manifestants sont bel et bien leurs premières victimes ; ... Oui ! ... de protection pour les journalistes, garants de notre liberté de savoir et de commenter, et qui ont été bien trop souvent lâchement attaqués ! ... de protection pour les commerçants, pour tous les Français, car les violences pèsent sur eux, détruisent leur travail et ruinent parfois les efforts d'une vie ; de protection pour les forces de l'ordre, aussi, qui accomplissent leur devoir et devraient pouvoir le faire en toute sécurité de protection pour la République, pour les élus, pour les institutions, que des petits groupes, de tout petits groupes d'ultra-violents croient pouvoir renverser. et peut-être plus que tout, c'est un texte de libertés : liberté de manifester sans crainte ; liberté de descendre dans la rue, d'exprimer des revendications, de faire entendre sa voix. Cette proposition de loi l'affirme haut et fort : il n'y a pas de place pour la peur dans les manifestations. Les événements des dernières semaines nous en ont rappelé l'urgence. Depuis le 27 novembre 2018, les brutes ont un bilan clair : environ 1 500 blessés parmi les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers.

C'est un choix de responsabilité. Oui ! Par cette décision, vous avez fait passer le sens de l'État, l'intérêt général, la protection des manifestants comme celle des forces de l'ordre avant toute position partisane. Vous avez montré que, face à des phénomènes graves, face à des violences durables, majorité et opposition étaient capables de travailler de concert. Lors de la première lecture, en octobre dernier, Laurent Nunez avait donné un avis de sagesse, approuvant les objectifs de cette proposition de loi, mais appelant à retravailler les dispositifs proposés.

et s'assurer qu'il dispose de tous les garde-fous nécessaires pour les libertés publiques. L'article 1 du texte permet, sur les lieux d'une manifestation ou à ses abords immédiats, et exclusivement sur réquisitions écrites du procureur de la République, de procéder à des fouilles de sacs et de confisquer toutes les armes ou les armes Personne, ici, n'est naïf : quand un individu vient dans une manifestation avec des boules de pétanque, ce n'est pas pour disputer une partie de pétanque, mais c'est bien pour blesser nos forces de l'ordre ou des manifestants. L'article 1, dans la rédaction que vous avez retenue en commission, permet d'intercepter de telles personnes avant qu'elles ne passent à l'acte. L'article 2 a fait couler beaucoup d'encre.

Ce texte ne comporte pas une once d'arbitraire. Au contraire, il prévoit toutes les précautions pour éviter le fait du prince. Chaque décision d'interdire de manifester doit être argumentée, motivée, proportionnée. Elle doit être directement liée à des comportements violents lors des manifestations. Ces dispositions ciblent précisément un petit nombre d'individus ultra-violents et ne peuvent, en aucun cas, dériver ou être généralisées. Non, il ne s'agit pas d'une proposition de loi liberticide. Au contraire, nous avons veillé, ensemble, à ce que la rédaction du texte protège les libertés. Le juge des référés

c'est, aujourd'hui, une possibilité dont dispose le préfet -, il cible ceux qui cassent et qui attaquent. Plutôt que de laisser faire, nous proposons d'empêcher quelques ultra-violents de manifester. Ainsi, nous permettons à tous de continuer à faire entendre leur voix.

Toutefois, cet article doit nous permettre d'agir rapidement : c'est son but. Or nous savons qu'une condamnation définitive peut prendre du temps. L'article 3 donne aux forces de l'ordre tous les outils pour contrôler les personnes interdites de manifester en les inscrivant, uniquement le temps de l'interdiction, sur le fichier des personnes recherchées. L'article 4 aggrave les sanctions en cas de dissimulation de son visage au cours ou à la fin d'une manifestation marquée par des troubles. Parmi les autres mesures de ce texte, les peines contre ceux qui détruisent sont renforcées, et une mesure juste, nécessaire, attendue est introduite : le principe du casseur-payeur. En effet, il est temps de mettre les vandales face à leurs responsabilités. Mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi est un texte de bon sens. La brutalisation au sein des manifestations n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui s'installe ; un phénomène qui, chaque samedi, depuis fin novembre, Forces de l'ordre, sapeurs-pompiers ou « gilets jaunes », près de 4 000 personnes ont été blessées depuis le 17 novembre dernier. Rien qu'à Paris près de 2 000 magasins ont été attaqués. C'est un bilan humain et matériel auquel nous ne pouvons pas nous habituer ; et c'est un bilan qui s'alourdit au fil des années de violences. en prononçant ces mots, je ne suis pas sourd aux appréhensions, aux craintes. Ah, « en même temps » ! Je les entends. Je suis convaincu par ce texte, mais j'estime qu'en matière de libertés publiques toutes les garanties doivent être prises.

Détourner le regard, c'est donner un laisser-détruire à quelques brutes. Qualifiez-les autrement ! Ne rien faire, c'est permettre à quelques ultra-violents de menacer nos vies, nos institutions et même notre liberté.

ce texte est l'occasion d'agir ; d'agir pour eux ; d'agir pour tous les Français ; une occasion à saisir pour tout responsable politique, pour tout républicain, pour tout protecteur des libertés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le depuis maintenant plusieurs mois, nous déplorons, semaine après semaine, en marge des manifestations organisées par le mouvement des « gilets jaunes », des dégradations dans nos centres-villes, des agressions contre des policiers ou des gendarmes, des magasins pillés, des voitures incendiées, du mobilier urbain détruit. Ces images choquent nos concitoyens, y compris ceux, nombreux, qui comprennent, voire approuvent les revendications défendues par ce mouvement social. Cela fait, à vrai dire, plusieurs années que les manifestations ont pris une tournure violente dans notre pays : on se souvient des violences commises à Nantes ou à Rennes dans le sillage du mouvement d'occupation de Notre-Dame-des-Landes de celles qui ont émaillé les mobilisations contre le projet de loi Travail en 2016 ; ou encore, l'an dernier, des violences des Black Blocs qui ont perturbé le traditionnel défilé syndical du 1 mai. Face à cette évolution de fond, nous voulons doter nos autorités administratives et judiciaires d'outils juridiques nouveaux pour les aider à garantir la tranquillité et la sécurité publiques, à laquelle aspirent nos concitoyens. C'est le but visé par la proposition de loi que nous examinons en deuxième lecture cette après-midi. Déposée par notre excellent collègue, le président Bruno Retailleau, ... Très bien ! ... et par plusieurs de nos collègues, elle a été adoptée par la Haute Assemblée le 23 octobre 2018, puis par l'Assemblée nationale le 5 février dernier. Je me réjouis que le Gouvernement, qui avait au départ exprimé des réserves sur ce texte, ait finalement décidé de le soutenir. Je ne peux que regretter cependant que tant de temps ait été perdu. Eh oui ! En effet, les dispositions de ce texte auraient été très utiles à nos forces de l'ordre au cours des derniers mois. Nous sommes tous, moi la première, profondément attachés au droit de manifester. Ce texte n'a pas et n'a jamais eu pour objectif d'entraver le droit de manifester il s'agit au contraire d'en garantir le libre exercice ... Tout à fait ! ... en ciblant un petit nombre de délinquants qui, par leurs actes violents, prennent en otage ceux de nos concitoyens qui défendent des revendications légitimes de justice sociale. de loi comporte un volet préventif, destiné à doter l'autorité administrative et nos forces de l'ordre de nouveaux outils pour prévenir les actes de violence et de dégradations commis dans le cadre des manifestations, et un volet répressif, pour permettre à l'autorité judiciaire d'apporter une réponse plus rapide et plus ferme aux auteurs de ces actes. Sur ces deux volets, l'Assemblée nationale a apporté des modifications destinées à rendre la proposition de sans toutefois remettre en cause les objectifs visés par le Sénat. S'agissant du volet préventif, l'Assemblée nationale a approuvé, dans leur principe, la plupart des dispositions que nous avions votées. L'article 1 adopté par le Sénat prévoyait de confier au préfet la possibilité d'instaurer des périmètres de contrôle aux abords des manifestations. Plutôt que de créer cette nouvelle mesure de police administrative, l'Assemblée nationale a préféré autoriser, sur réquisitions du procureur de la République, des fouilles de sacs et de véhicules, afin d'éviter l'introduction d'armes dans les manifestations. Les représentants des forces de l'ordre que j'ai reçus en audition ont estimé que cette mesure répondrait efficacement à leurs besoins sur le terrain. Malgré quelques réticences initiales, l'Assemblée nationale a également souscrit à l'article 2, qui prévoit la création d'une mesure d'interdiction administrative de participer à une manifestation. Le Sénat avait été très attentif à entourer cette mesure de suffisamment de garanties. Je me félicite de ce que les députés les aient conservées, en particulier pour ce qui concerne le droit au recours effectif. Afin de répondre aux besoins du terrain, l'Assemblée nationale a élargi le périmètre de la mesure : l'interdiction de manifester pourra concerner non seulement des personnes ayant commis un ou plusieurs actes violents à l'occasion de précédentes manifestations, y compris lorsqu'elles n'ont pas encore été condamnées, mais aussi des personnes qui constituent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en raison de leurs « agissements » à l'occasion de précédentes manifestations. En outre, les députés ont prévu la possibilité, pour le préfet, de prononcer des interdictions de manifester valables sur l'ensemble du territoire, pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsque la personne concernée est susceptible de participer à plusieurs manifestations concomitantes sur le territoire ou successives dans le temps. La commission s'est demandée si, avec cet élargissement, la mesure conservait un caractère suffisamment proportionné, au regard de ses effets potentiels sur l'exercice du droit de manifester et de la liberté d'aller et venir. Mes chers collègues, il nous a été assuré que son application serait très ciblée. Seules les personnes les plus dangereuses seraient concernées, quelques dizaines à Paris, tout au plus quelques centaines sur l'ensemble du territoire. Il s'agit bien de tenir à l'écart de la manifestation les « casseurs », qui ont pour seul objectif de causer des dégâts. En tout état de cause, les arrêtés d'interdiction seront soumis au contrôle du juge administratif, qui s'assurera, comme pour toute mesure de police administrative, de leur caractère nécessaire et proportionné. S'agissant de l'article 3, l'Assemblée nationale a estimé préférable d'inscrire les mesures d'interdiction de manifester dans le fichier des personnes recherchées, document aisément consultable par les forces de police et de gendarmerie, plutôt que de créer un nouveau fichier. Il s'agit, à nos yeux, d'une mesure de simplification bienvenue. les députés ont complété ce volet préventif par deux articles additionnels, qui ne soulèvent vraiment pas de difficulté : le premier vise à assouplir les modalités de déclaration des manifestations auprès de l'autorité administrative ; le second prévoit un contrôle parlementaire renforcé, notamment avec la remise d'un rapport annuel au Parlement. S'agissant, à présent, du volet répressif, je m'attarderai surtout sur l'article 4, relatif à la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation. En octobre dernier, nous avions soutenu la création de ce délit, qui présente de réels avantages sur le plan opérationnel : elle permettra l'interpellation et le placement en garde à vue de personnes qui dissimulent leur visage. En première lecture, notre commission avait veillé à bien caractériser l'élément intentionnel du délit, en précisant que la dissimulation du visage devait avoir pour objectif de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des troubles à l'ordre public. Redoutant que cet élément ne soit difficile à établir devant les tribunaux, l'Assemblée nationale a retenu une rédaction plus concise. Elle met l'accent sur l'existence ou non d'un motif légitime de se couvrir le visage. de se couvrir le visage. Je l'avoue, nous nous sommes demandé si cette définition était satisfaisante au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, qui impose de définir avec précision tous les éléments constitutifs d'une infraction pénale. d'une infraction pénale. Toutefois, les représentants du ministère de l'intérieur comme de la Chancellerie que nous avons entendus ont estimé que cette rédaction était acceptable, étant précisé qu'il appartiendra au parquet d'établir devant le tribunal correctionnel que la personne mise en cause n'avait pas de raison légitime de se couvrir le visage. En matière pénale- je vous le rappelle -, la charge de la preuve ne saurait reposer sur la personne mise en cause. Compte tenu de ces assurances, notre commission a décidé de s'en tenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, afin de doter rapidement nos forces de l'ordre d'un outil qui leur sera très utile pour extraire d'une manifestation des éléments perturbateurs. La commission des lois a ensuite confirmé la suppression de l'article 5, relatif au port d'arme et au jet de projectile, considérant que ses dispositions étaient satisfaites par les textes et par la jurisprudence en vigueur. elle a approuvé les modifications introduites à l'article 6, relatif à la peine complémentaire d'interdiction de manifester, ainsi qu'à l'article 7, relatif à la mise en cause de la responsabilité civile des auteurs de dommages lors d'une manifestation. Au total, en dépit des interrogations que j'ai mentionnées, notre commission a choisi d'adopter la proposition de loi sans modification. Des garanties importantes m'ont été apportées, tant par le ministère de l'intérieur que par la Chancellerie, quant au travail mené par leurs services pour garantir un juste équilibre entre efficacité des mesures et respect des droits et libertés. Le Président de la République a annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel : ce dernier aura donc l'occasion de se prononcer sur le texte. Dans le contexte actuel, les interrogations sur la proportionnalité de certaines dispositions ne doivent pas nous faire oublier les nombreuses garanties apportées au texte. Je crois surtout qu'il nous revient, en tant que législateur, de faire preuve de responsabilité, en dotant nos forces de l'ordre des moyens nécessaires à la prévention des violences. Il s'agit non seulement d'assurer la sécurité de nos concitoyens, mais de garantir le libre exercice du droit de manifester je vous remercie

Inspiré de la loi anti-casseurs de 1970, ce texte a très vite provoqué des réactions mitigées. Partiellement épurée en commission, sa rédaction restait, de l'avis général, perfectible. Elle a beaucoup évolué à l'Assemblée nationale.

Disons-le clairement : oui, ce texte présente un risque d'arbitraire. Mais non ! En définitive, il peut permettre au préfet, donc au Gouvernement, de choisir ses manifestants. Pour des raisons de fond et de forme que je vais vous détailler, je ne vois pas d'autre solution pour notre assemblée que d'interrompre, ici, le cheminement législatif de cette proposition de loi. Commençons par la forme. Alors qu'il s'agissait d'un texte relatif aux libertés publiques, la majorité sénatoriale avait fait le choix d'une proposition de loi. En évitant ainsi toute étude d'impact et toute consultation de grande envergure, les élus du groupe Les Nous avions souligné ce manque de concertation en première lecture. Depuis cet automne, la concertation a en quelque sorte eu lieu : on ne compte plus les prises de position hostiles à ce texte, que ce soit dans les rangs des syndicats,

Ce sont MM. Sureau et Mignard, soutiens d'Emmanuel Macron, qui prennent bruyamment leurs distances. L'absence de consultation initiale était compréhensible, s'agissant d'une initiative portée par un groupe politique. Mais cette méthode est devenue beaucoup plus problématique dès lors que le Gouvernement a décidé de reprendre à son compte cette proposition de loi. Avec le lifting des amendements gouvernementaux, ce texte a changé de nature, mais la mue n'a pas été complètement opérée. Faisons-nous face à un texte porté par la droite ? Par les macronistes ? Par les deux ? La République En Marche n'a pas souhaité l'assumer jusqu'au bout, et cela s'est senti dans les hésitations observées à l'Assemblée nationale et au Gouvernement. Le Gouvernement et la majorité des députés sont-ils satisfaits par ce texte qu'ils ont réécrit ? On ne sait plus ! Des députés voulaient voter contre, mais ils se sont abstenus, parce que le texte qu'ils venaient de réécrire allait de nouveau être réécrit. de la majorité sénatoriale, ce n'est guère plus clair. Chers collègues, vous avez d'abord dénoncé la réécriture du texte, en laissant entendre que vous alliez le corriger. Finalement, vous ne corrigez rien, préférant faire un pari de Pascal revisité. Si le Conseil constitutionnel existe et censure ce texte, vous aurez beau jeu de dénoncer le mauvais travail des députés. En revanche, si le Conseil constitutionnel se fait oublier, vous revendiquerez la paternité de cette loi

l'Élysée va-t-il saisir les Sages à propos des articles 2, 3 et 6 ... On a connu mieux comme reconnaissance de paternité ! Cette proposition de loi Retailleau-Castaner-Macron se retrouve orpheline. Et pourtant, elle prend le chemin d'une adoption conforme Sur le fond, les arguments en défaveur du texte qui nous est proposé aujourd'hui ne manquent pas. Notons, d'abord, que celui-ci puise son inspiration dans l'arsenal anti-hooligans. Cet arsenal est-il toutefois si parfait qu'il puisse être généralisé ? On ne le sait pas, parce qu'il n'a jamais été évalué. À vrai dire, on a bien une petite idée de la pertinence de ce dispositif et des interdictions administratives de stade, les IAS. Il faut écouter l'Association nationale des supporters, qui dénonce les actes de violence, mais prend la défense des supporters victimes des des mailles d'un filet mal pensé. On découvre ainsi des histoires absurdes de supporters blanchis par la justice pénale, mais qui doivent continuer à batailler devant la justice administrative pour faire lever une IAS prononcée contre la mauvaise personne.

Monsieur le ministre, pourriez-vous informer la représentation nationale des évaluations qui doivent être faites des interdictions administratives de stade ? Proposition de loi orpheline, mal inspirée, cette loi anti-manifestants est aussi, si ce n'est surtout, dangereuse pour les libertés publiques. Elle contient un grand nombre de dispositions qui se révéleraient extrêmement risquées si elles se retrouvaient entre les mains d'un parti non républicain. Pire, elle pourrait même donner de mauvaises idées à un parti républicain. Ainsi, l'article 2 crée une interdiction administrative de manifester dans une version plus répressive que la version sénatoriale. Selon nous, cet article porte atteinte à la liberté d'expression collective des opinions et à la liberté d'aller et venir, en raison du pointage en commissariat, déjà évoqué. Bien qu'elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation, par le représentant de l'État dans le département ou par le préfet de police, d'agissements doublés d'un risque supposé de « menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » et,, pourrait s'appliquer à des manifestations non déclarées « dont [le représentant Faute d'énoncer des critères suffisamment précis et restrictifs, la décision d'interdiction préventive de manifester sera laissée à la seule appréciation du préfet. Les garde-fous prévus dans le texte à l'article 2 présentent un caractère formel : dans certains cas, l'arrêté du préfet serait « exécutoire d'office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation En d'autres termes, le droit à un recours effectif devant le juge sera rendu impossible dans les faits. L'article 4 de la proposition de loi crée un délit passible d'une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour dissimulation du visage dans une manifestation. À la suite des travaux du Sénat visant à caractériser l'intentionnalité du délit, Mme Alice Thourot, rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait souhaité apporter encore plus de précisions,

L'article 4 de la proposition de loi viserait ainsi, outre des personnes qui se trouveraient « au sein » de la manifestation, des personnes qui seraient à ses « abords immédiats », alors que des troubles à l'ordre public ne sont pas pas en train d'être commis, mais « risquent d'être commis », sans qu'un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimulerait seulement une « partie de son visage Pour que la loi qui impose une restriction à ses droits garantis soit accessible au citoyen, celle-ci doit être précise et prévisible, de sorte que celui-ci soit en mesure de connaître la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision est le corollaire du principe de sécurité juridique. Elle est inhérente à l'objectif d'intelligibilité de la loi. J'ai, pour ma part, du mal à imaginer ce que recouvriraient en pratique, sur le terrain, les « abords immédiats » d'un parcours Bastille-République. L'article 6 a été inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à la faveur d'un amendement de sa rapporteure adopté au stade de l'examen du texte en commission des lois. Il complète la liste des obligations et des interdictions auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Il y ajoute notamment l'interdiction de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention. Or, dans le droit en vigueur, le contrôle judiciaire peut d'ores et déjà comporter l'interdiction, pour le mis en cause, de se rendre dans certains lieux. L'article 6 est donc superflu. Par cette motion, notre groupe souhaite attirer l'attention du plus grand nombre de sénateurs sur les risques que ce texte comporte. En première lecture, de nombreux collègues de la majorité présidentielle avaient assumé leur choix et marqué leur opposition à ce texte. Nous leur donnons aujourd'hui l'occasion de réitérer cette affirmation de leurs convictions. Le nombre de personnes interpellées au cours des manifestations récentes comme la lourdeur des peines prononcées en comparution immédiate indiquent que des réponses juridiques existent déjà. Je vous demande très solennellement, mes chers collègues, que nous assumions, que le Sénat assume son rôle de gardien des libertés publiques. Épargnons-nous ce texte inutile, imprécis et dangereux.

affirme que, jamais, le préfet ne pourra remplacer le juge

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite évoquer devant vous l'origine de ce texte. Je fus témoin de violence politique pendant des années, bien avant novembre 2018, 2018, notamment lors des manifestations contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les centres-villes de Nantes et de Rennes furent régulièrement dévastés et vandalisés par des groupes de casseurs ultra-violents et très organisés. Ces faits s'étalèrent sur de nombreuses années. Antérieurement à ces années-là, je fus également victime de cette violence politique, poussée à son paroxysme. Je vous précise d'ailleurs que, le 15 novembre dernier, j'ai été amené à faire un signalement auprès du procureur de la République pour de nouvelles menaces de mort. Je vais vous narrer un événement qui remonte au 24 novembre 2000. À La Baule, un colis piégé explosait au siège du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise, dont j'étais alors président,

Après plusieurs mois d'une enquête rigoureuse menée par la police judiciaire de Nantes, que je remercie encore de son professionnalisme et de son abnégation, trois personnes furent arrêtées. Un quatrième complice avait disparu, éliminé physiquement par les trois autres. Ce groupe de militants d'extrême droite avait des relents néonazis. Il y eut trois procès d'assises, le premier à Nantes, le procès en appel à Rennes et un troisième à Versailles, l'assassinat de leur complice ayant été dissocié de l'attentat au colis piégé. cinq longues journées. J'ai assisté, en ces instants, chez les policiers, chez les magistrats, chez les jurés populaires à la recherche de la vérité, parfois au confluent de la présomption d'innocence et de l'intime conviction. La phrase qui m'a le plus marqué, lors de ces longues semaines d'audience, a été prononcée par le principal accusé, reconnu coupable, qui avouera être le commanditaire du colis piégé

qui savent que, pour renverser la démocratie fragile, des conditions exceptionnelles sont nécessaires, qu'il faut créer par la violence. Regardons l'histoire du XX siècle, du fascisme au nazisme, des Brigades rouges à la bande à Baader, en passant par Action directe, pour nous en instruire.

Vous vivez avec le remords de la chance coupable, avec à la fois la satisfaction du triomphe de la vérité et le cours des choses irréversibles, car on ne fait pas revenir à la vie à la vie les morts d'aujourd'hui et d'hier. De même, si l'on peut réparer les vivants, ce n'est souvent que partiellement. Les mutilations taraudent traditionnellement et quotidiennement, tant physiquement que psychologiquement, ceux qui en sont victimes.

une majorité qui tutoyait l'unanimité -, je me suis levé pour faire une ovation debout au meilleur des orateurs de cette journée historique, celui qui fut garde des sceaux, notre collègue au Sénat, qui était, ce jour-là, le porte-parole du groupe du parti socialiste : M. Robert Badinter. Mes chers collègues, de loi n'est en rien liberticide. Nous nous opposons à cette motion, car l'âme de ce texte, c'est l'esprit de la République, cette République une et indivisible, la République des droits et devoirs, cette République au triptyque que le monde entier nous a emprunté à chaque fois que l'on voulait faire émerger et faire vivre la démocratie, ces trois mots sculptés sur le fronton de nos bâtiments républicains et qui résonnent plus encore aujourd'hui, dans cet hémicycle : la liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la République, vive la France

Les interrogations soulevées par les auteurs de la motion sont légitimes, mais ne doivent pas nous conduire à remettre en cause le bien-fondé et l'utilité des dispositions de ce texte. Nous avons aujourd'hui besoin de nouveaux outils pour pour prévenir l'infiltration dans les manifestations de personnes dont l'unique objectif est de commettre des violences à l'encontre de nos institutions, de nos symboles et de nos forces de l'ordre. Ce texte n'a pas, et n'a jamais eu, pour objet de porter atteinte au droit de manifester. Ne nous méprenons pas : ceux qui, depuis plusieurs semaines, nuisent à l'exercice du droit de manifester, ce ne sont ni les autorités ni les forces de l'ordre, mais bien les casseurs Cette proposition de loi vise uniquement à empêcher que ces individus, je dirais même ces délinquants, infiltrent les manifestations et prennent en otage des citoyens qui souhaitent exprimer pacifiquement leurs revendications. Les mesures qu'elle contient ne sont pas soumises à l'arbitraire. Comme toute mesure de police administrative, elles devront être mises en oeuvre dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Chacune d'entre elles sera soumise au contrôle du juge administratif, qui, je le rappelle, a démontré, au cours des dernières années, son rôle de protecteur des libertés.

de l'ordre public imposé par l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est manifestement rompu, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce

l'article X du texte fondateur de 1789. L'addition des articles, à l'exception du modeste article 1 A, porte gravement atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, dont le véhicule est, justement, le droit de manifester. L'article 2, en transférant à l'autorité politique le pouvoir d'interdire à une personne de manifester, de surcroît, sur l'ensemble du territoire et pour une durée maximum d'un mois, ne pourra qu'être jugé non conforme à la Constitution. C'est inéluctable ! L'article 4, qui sanctionne lourdement la dissimulation du visage, même partielle et sans élément intentionnel, ne respecte pas non plus les libertés fondamentales. L'article 6, sur les peines complémentaires, pose également de lourdes questions. Les modifications apportées par la majorité de l'Assemblée nationale au texte sénatorial ont provoqué un dérapage incontrôlé la décision d'Emmanuel Macron de saisir lui-même le Conseil constitutionnel se rapproche de la sortie de route. Le Président de la République est piégé par un texte de circonstance,

que mon groupe souhaite s'associer à la saisine du Conseil constitutionnel qui est en cours de préparation, en rappelant que soixante sénatrices et sénateurs peuvent exercer ce droit.

Dans cet hémicycle où le respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs est un principe important, que nous avons dû défendre encore récemment, je ne peux m'empêcher de revenir sur deux points.

J'ose espérer, mes chers collègues, que, lorsque cela se produira dans d'autres circonstances, vous saurez rappeler aux membres du Gouvernement l'attitude qu'ils doivent adopter

Si je reviens sur ce dernier point, c'est qu'il se dit des choses inexactes. On prétend que ce texte permet l'accès au juge, car, dans le cadre du référé-liberté, le juge administratif peut être saisi.

qui s'intègrent dans les cortèges pour les dévoyer, qui menacent le droit de manifestation, qui pratiquent systématiquement les violences contre nos forces de l'ordre

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.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

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Je suis saisi, par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste,

monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, « avec cette loi, on transfère aux préfets des pouvoirs que détiennent les juges. [ ...] Nous touchons donc à l'État de droit, et c'est proprement inacceptable Ces mots, mes chers collègues, n'émanent pas d'un dangereux agitateur, mais sont ceux de Charles Amédée de Courson, député centriste de la Marne, connu pour ses convictions libérales sur le plan économique. Nous nous retrouvons aujourd'hui, avec des hommes et des femmes d'horizon très divers, pour combattre une proposition de loi qui porte gravement atteinte à plusieurs libertés constitutionnelles, à commencer par le droit de manifester. C'est le 7 janvier 2019 qu'Édouard Philippe, très martial, a annoncé sa volonté de reprendre pour le compte du Gouvernement la proposition de loi adoptée par le Sénat le 23 octobre 2018, trois semaines avant la première manifestation des « gilets jaunes », le 17 novembre. Le changement d'attitude du Gouvernement par rapport à ce texte est manifeste : M. Nunez citait en octobre l'article de la Déclaration des droits de l'homme fondant le droit de manifester et recommandait d'attendre et de bien réfléchir avant de légiférer

ont tenté d'étouffer les revendications du mouvement des « gilets jaunes » par la mise en exergue d'actes violents, spectaculaires, qui sont le fait d'une infime minorité de manifestants. Monsieur le ministre, je l'ai dit et répété le 7 mars dernier, lors de l'examen de notre proposition de loi visant à interdire les LBD 40 : les fonctionnaires de police ne sont pas responsables collectivement de la situation actuelle. Vous les envoyez en première ligne, avec des ordres et une doctrine qui ne permettent pas l'apaisement. Notre opposition à ce texte, à la stratégie de la tension mise en oeuvre, vise à protéger autant les policiers que les manifestants Comment ne pas faire le lien entre les mesures envisagées, sur lesquelles je reviendrai avant que mon amie Esther Benbassa ne les détaille dans la discussion générale, et ces propos dangereux, d'une responsabilité mal assurée, d'Emmanuel Macron : « il il faut maintenant dire que, lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire » ? Avec ces propos, M. Macron ne calme pas le jeu ; il souffle sur les braises, espérant, comme nombre de ses prédécesseurs, que la provocation à la violence permettra un pourrissement du mouvement. Face à la persistance du soutien de l'opinion et des manifestations, malgré les difficultés d'exercer ce droit constitutionnel, le Président de la République devrait plutôt regarder la vérité en face seule une réponse politique aux aspirations populaires portées par ce mouvement et profondément ancrées dans les villes et les campagnes, seule une réponse politique à cette formidable exigence de dignité et de démocratie, seule une réponse politique aux salariés et aux retraités qui demandent tout simplement à vivre, qui attendent une nouvelle répartition des richesses assurant l'égalité, seule cette réponse politique permettra de résoudre cette crise ! Monsieur le ministre, par le passé, seule une réponse politique a permis de dénouer des crises qui, elles aussi, comportaient, comme tout soulèvement populaire, leur part de violence. Depuis sa présentation, puis son adoption à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi suscite un véritable tollé. Comment ne pas rappeler les propos de M. Toubon ? Il l'estime « déséquilibrée, attentatoire aux libertés et susceptible d'exposer les forces de l'ordre à davantage de risques et de dégrader leur relation avec la population En cela, M. Toubon est fidèle aux valeurs d'une droite républicaine qui sait que l'usage disproportionné de la force met en danger l'équilibre de la société.

Frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. [ ...] Il est encore plus grave de frapper des manifestants après leur arrestation. [ ...] Dites-vous bien et répétez-le autour de vous toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de camarades qui souhaitent se venger. Cette escalade n'a pas de limites. » Voilà les propos du préfet Grimaud ! Eh oui ! Oui, monsieur le ministre, votre choix de l'escalade constitue un danger démocratique. associations et syndicats l'affirment : « Cette loi de circonstance porte un lourd risque d'arbitraire des gouvernements d'aujourd'hui comme de demain. Les violences contre les personnes, les biens, les institutions qui ont eu lieu ne peuvent justifier qu'un exécutif s'arroge des pouvoirs exorbitants et décrète qui peut ou ne peut pas manifester. » Il ne s'agit pas de cela ! Oui, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi met en péril la liberté de manifester quelques remarques sur les points essentiels de ce texte. L'article 2, qui, dès l'origine sénatoriale, transférait le pouvoir d'interdire à une personne de manifester du juge au préfet, c'est-à-dire au représentant du pouvoir politique, courait le risque d'inconstitutionnalité au point, comme le reconnaît le président Bas, de devoir être strictement encadré. D'ailleurs, le Président de la République lui-même s'interroge, puisqu'il a annoncé, hier, vouloir saisir le Conseil constitutionnel. on marche sur la tête : pourquoi le Président de la République annonce-t-il, la veille du débat sénatorial, la saisine du Conseil constitutionnel, alors que le Sénat s'apprête à voter conforme ce texte, si la majorité Les Républicains le vote ainsi ? À l'Assemblée nationale, plus de faux-semblants ni de préventions : l'article 2 a été musclé au point de prévoir que l'interdiction puisse être assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de manifester sur tout le territoire, pour une durée pouvant De plus, les députés ont décidé que les personnes interdites pourraient ne pas avoir été condamnées préalablement et pourraient n'avoir commis que des « agissements » durant un rassemblement précédent- terme vague, inspiré de la loi anti-hooligans. Mais, monsieur le ministre, mes chers collègues, supporter une équipe, ce n'est pas exercer un droit constitutionnel ! Cet élargissement important du champ de l'article 2 expose celui-ci à une censure, comme il a été souligné lors des interventions sur la motion d'irrecevabilité. D'ailleurs, Mme la rapporteure a rappelé ce danger, tout comme le président de la commission des lois, devant la presse et en commission. Hier, donc, c'est M. Macron qui a annoncé sa volonté de saisir le Conseil constitutionnel, sans doute pour faire bonne figure. Pourquoi le législateur ne prend-il pas ses responsabilités ? Pourquoi renvoyer cette mission au Conseil constitutionnel, dont, je le rappelle, la légitimité n'est pas la même que celle des assemblées républicaines ? L'article 3, qui concerne le fichage- un de plus ... -des personnes interdites de manifestation, porte également atteinte aux libertés individuelles, d'autant que l'Assemblée nationale entend mêler dans un même fichier

selon vos souhaits, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, il s'expose aussi, selon Mme la rapporteure, à l'inconstitutionnalité, l'Assemblée nationale ayant supprimé, sur l'initiative d'un député En Marche, Mme Laurence Vichnievsky, l'élément intentionnel. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons constaté l'utilisation massive de gaz lacrymogènes durant les manifestations, déclarées ou non. Lors de certains rassemblements, des milliers de grenades ont été utilisées. Comment oser empêcher un manifestant de se protéger ? Si l'élément intentionnel est supprimé, même les personnes tentant de protéger leur respiration seront visées et ne pourront exercer le droit constitutionnel de manifester ! Pour vous dire

si une trace doit rester dans l'histoire de ce mouvement, outre son originalité, sa force, sa persistance et, ne vous en déplaise, sa popularité, c'est la répression systématique et violente qui s'abat sur lui. Après le Défenseur des droits, le Conseil de l'Europe, l'ONU même, ce sont trente-cinq ophtalmologistes, professeurs de renommée internationale, qui ont écrit à Emmanuel Macron pour demander un moratoire ... Sur les manifestations ? ... sur l'utilisation des LBD 40. Il faut aujourd'hui interdire cette arme Mes chers collègues, ce nouveau monde est étonnant : il reprend à son compte une vieille loi adoptée en 1970, la loi anti-casseurs. Faire du vieux avec du vieux pourrait être leur doctrine, votre doctrine, monsieur le ministre ne changez pas de cap, mais, pour tenter désespérément de le maintenir, vous vous appuyez sur la répression ! Le vote conforme proposé au Sénat, qui vole au secours d'Emmanuel Macron en la matière, vise à contrer l'impopularité croissante de la politique répressive, y compris au sein de la majorité. précipitation est un aveu de faiblesse. Les valeurs profondes de notre République, qui ont marqué l'histoire de notre pays, malgré les tragédies et les souffrances, s'imposeront, j'en suis certaine. Le Sénat, qui s'affirme comme le gardien des libertés, n'a qu'une chose à faire pour ne pas trahir sa parole : rejeter d'emblée ce texte, dire « stop

... L'ordre républicain, c'est un partage entre la liberté, la démocratie, la sécurité, la République.

La République s'est régulièrement défendue, et la République doit se défendre. La liberté est un droit ; manifester est un droit ; l'équilibre est un droit. Mais de quoi, de qui, parle-t-on ? Aujourd'hui, monsieur le ministre, l'armée de la République, la gendarmerie de la République, la police de la République

à des gens qui ne respectent pas la démocratie, qui ne veulent pas de la République et qui, non seulement en France mais partout en Europe, remettent en cause les systèmes démocratiques.

de la République et de la démocratie, à part des contestations et des colloques ? Que faisons-nous, en réalité, devant cette évolution, inéluctable, de la violence, de la remise en cause des droits et des libertés ? Alors oui, la République doit se défendre. Oui, naturellement, la démocratie n'existe que si elle se défend. Je ne suis pas- je l'ai toujours dit -un adepte des comparaisons avec les années trente, parce que les conditions politiques, économiques, militaires, internationales de l'époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Mais, tout de même,

: donnez aux forces de l'ordre, aux forces de l'ordre de la République, aux autorités légitimes de la République, les moyens de faire en sorte

contesté par une petite minorité, qui profite de toutes les manifestations, d'où qu'elles viennent, pour remettre en cause la République et la démocratie. Alors oui,

ce n'est plus la situation d'aujourd'hui, et pas seulement en France. Pourquoi ? Voyez ce qui se passe partout en Europe, et même dans le monde : partout, les minorités violentes ont décidé de profiter des grandes manifestations, des manifestations de masse, pour déstabiliser la démocratie et la République.

où les forces de sécurité, les autorités légitimes de la République, le Parlement ont besoin que chacun soit dans son rôle, assume et incarne.

avec ce que cela veut dire, défendre la République, la démocratie dans notre pays ? Il faut les défendre

Face aux violences, aux dégradations, notre responsabilité de législateur est de doter rapidement nos forces de l'ordre de tous les moyens nécessaires pour garantir tant la liberté de manifester que la sécurité de nos concitoyens. Pouvons-nous encore tolérer que, chaque samedi, nos centres urbains soient saccagés par les pilleurs ? Pouvons-nous accepter que nos forces de l'ordre continuent, chaque semaine, d'être la cible de jets de pavés, de boules de pétanque et de bouteilles d'acide ?

ne se refusera à applaudir les forces de l'ordre ou l'armée. Seulement, il ne suffit pas de convoquer la République et ses forces de l'ordre légitimes pour avoir raison sur le fond ! Ce texte est déséquilibré

ensuite parce qu'il entend s'adapter à la situation actuelle, dans laquelle nos forces de l'ordre subissent des violences et des attaques absolument inacceptables dans notre République.

Je disais donc que je suis contre ce texte, mais que je ne l'aurais pas été je ne l'aurais pas été s'il était accompagné ou s'il avait été précédé de mesures de fond pour essayer de répondre au malaise social qui monte depuis des années, non seulement en France, comme l'a souligné Roger Karoutchi, dans l'Europe entière. On nous bassine avec la menace de l'extrême droite, mais vous fabriquez des électeurs d'extrême droite tous les jours,

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, il est des questions qu'on ne peut aborder sans un profond découragement et sans une amère tristesse ». Ainsi Benjamin Constant commençait-il son discours à la Chambre des députés, le 7 mars 1820. Découragement oui, tristesse aussi, surprise assurément. Car, à l'évidence, personne n'imaginait, le 23 octobre dernier, lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture, ici, au Sénat, ce qu'il pourrait advenir de ce texte.

La crise des « gilets jaunes », ultérieure, a conduit le Gouvernement à se saisir de ce texte d'origine sénatoriale, ce qu'il n'aurait sûrement pas fait en d'autres circonstances. Dès lors, je considère, comme une partie des membres de mon groupe, que ce texte a changé de nature : il a basculé dans la catégorie des lois dites de circonstance, réaction politique à une crise qui envahit le débat public depuis plusieurs mois. Or nous devons être précautionneux, nous sénateurs plus que les autres, face au diktat de l'actualité ou face à une quelconque pression. Les circonstances politiques de notre vote d'aujourd'hui sont d'ailleurs différentes de celles du dépôt du texte. C'est pour moi une évidence. Le débat à l'Assemblée nationale a été enflammé : il a pu donner lieu à certains excès, tant chez les opposants à ce texte que chez ses partisans. Il a, par certains aspects, permis de mettre en lumière des questions qui restent devant nous. Une chose est sûre : le texte qui revient du Palais Bourbon n'est pas le même que celui qui a été adopté par le Sénat en octobre dernier. Je veux l'affirmer avec force et clarté, notamment à l'égard de notre collègue auteur de la proposition de loi, le président Bruno Retailleau.

brièvement sur les plus importantes. L'article 4 prévoit la création d'un délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation. Cette pratique est réprimée depuis 2009, mais par une simple contravention. basculer du domaine contraventionnel au domaine délictuel, le texte a une conséquence pratique immédiate : il rend possibles l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de l'infraction, aujourd'hui impossibles. L'intérêt est donc évident, et les modifications introduites par l'Assemblée nationale paraissent pertinentes, puisque nos collègues députés ont précisé l'élément intentionnel de cette infraction, afin de se conformer au principe de légalité des délits et des peines. De même, la modification introduite à l'article 3 nous semble pertinente, puisqu'elle évite la création d'un fichier en prévoyant une insertion dans le fichier des personnes recherchées. Voilà, mes chers collègues, pour les points positifs ... Reste l'article 2, qui prévoit l'interdiction administrative de manifester. Nous étions déjà réservés sur ce point en première lecture. Les modifications introduites par la majorité à l'Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, nous inquiètent nous inquiètent au regard de l'idée que nous nous faisons des libertés publiques dans notre pays. Elles nous inquiètent aussi par les imprécisions de rédaction qu'elles introduisent dans cet article 2.

mais, surtout, il prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire à une personne de manifester, cette interdiction pouvant aller jusqu'à un mois sur tout le territoire national. La question la plus sensible porte sur le fait de savoir sur quelle base les préfets vont pouvoir justifier une telle interdiction. En raison d'une condamnation pénale, pour des atteintes aux biens ou personnes ? Mais non Ils pourront interdire une personne de manifester pendant un mois pour des « agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ». C'est très bien ! Pouvait-on trouver formulation plus vague ou plus difficile à définir ? Et, surtout, les agissements en question auront-ils été soumis à l'appréciation d'un magistrat judiciaire ? Évidemment non Vous l'aurez compris, monsieur le ministre de l'intérieur, je suis profondément hostile, comme certains collègues de mon groupe, à cette disposition telle qu'elle a été rédigée et votée par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par le Sénat était profondément différent puisqu'il faisait, lui, référence à une condamnation pénale préalable. Eh oui ! La qualité du travail de notre rapporteure, Catherine Troendlé, que je tiens à saluer, a malgré tout permis de convaincre une majorité de membres de mon groupe. Ceux-ci sont parvenus à surmonter les craintes suscitées par cet article 2, étant convaincus que l'urgence de la situation impose au Sénat d'adopter définitivement ce texte aujourd'hui, mais ce n'est pas mon cas. Comme plusieurs de mes collègues, je ne peux pas voter cette proposition de loi en l'état. Notre rapporteure exprimait en première lecture sa volonté d'assurer, pour l'ensemble du texte, une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la protection

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, le droit de manifester, garanti par l'article VII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, semble aujourd'hui menacé. Dégradations de bâtiments institutionnels, de mobilier urbain, de bâtiments commerciaux ; destructions d'équipements publicitaires ; incendies de voitures ; jets de projectiles contre les forces de l'ordre ; CRS pris au milieu des flammes ; policiers blessés, frappés à terre Les actes de violence et de dégradation dans les manifestations deviennent récurrents. Ceux-ci ont pris une ampleur sans précédent : depuis le printemps 2016 et, plus récemment, depuis novembre dernier, chaque samedi, des groupes de « casseurs » sèment le trouble et s'en prennent, avec une violence inédite, à nos forces de l'ordre. Je fais ici référence aux récents événements qui ont fait la « une » de l'actualité, comme le saccage du musée de l'Arc de Triomphe, le pillage de commerces ou encore l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. Ces actes violents et inadmissibles, que l'on constate aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les villes moyennes, témoignent de l'urgence à équiper nos forces de l'ordre d'outils leur permettant de mieux les prévenir et de doter l'autorité judiciaire de dispositions, afin de les sanctionner plus sévèrement.

Le contexte inédit de ces dernières semaines confirme que cette proposition de loi comporte des dispositifs pertinents et utiles. Celle-ci contient en effet un volet préventif, qui tend à doter l'autorité administrative de nouvelles prérogatives pour mieux prévenir les débordements, ainsi qu'un volet répressif, qui vise à donner à l'autorité judiciaire les moyens de réprimer plus efficacement les violences et les actes de dégradation. le premier volet, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les objectifs visés par le Sénat, tout en apportant des modifications. Elle a notamment confirmé la possibilité donnée à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge des référés, d'interdire, par arrêté, à un individu de participer à une manifestation, si celui-ci constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Allant plus loin que ce que le Sénat avait prévu en première lecture, elle a, de plus, autorisé l'autorité administrative à interdire à un individu de prendre part à toute manifestation sur le territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois. Par ailleurs, elle a préféré, dans un souci de simplification, l'inscription de l'ensemble des mesures d'interdiction de manifester au sein d'un fichier existant : le fichier des personnes recherchées. Quant au second volet- le volet répressif -, l'Assemblée nationale a retenu une nouvelle définition du délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords d'une manifestation publique, qu'elle a jugée plus opérationnelle que la rédaction adoptée par le Sénat. En outre, elle a supprimé l'article relatif aux délits de port d'arme et de jets de projectiles, considérant que ces dispositions étaient satisfaites par le droit en vigueur. Elle a également complété les mesures approuvées par le Sénat concernant la peine complémentaire d'interdiction de manifester, en prévoyant la possibilité de recourir aux procédures rapides pour les délits liés à un attroupement, ainsi que la possibilité d'interdire à un individu de manifester en des lieux déterminés dans le cadre d'un contrôle judiciaire. l'Assemblée nationale a souhaité alléger le régime de déclaration des manifestations dans un nouvel article et a confirmé, sous réserve de quelques ajustements, le dispositif proposé par le Sénat concernant la responsabilité civile des auteurs de dommages. La plupart de ces modifications permettront de faciliter la mise en oeuvre par nos forces de sécurité et par l'autorité judiciaire des mesures nouvelles prévues par le texte. Monsieur le ministre, mes chers collègues, figurant dans cette proposition de loi visent bien à assurer le libre exercice du droit de manifester. Elles ne restreignent en rien les droits et libertés des manifestants, mais, au contraire, elles ciblent ceux qui, par leurs actes violents, prennent prennent en otage les manifestations et les rassemblements. L'évolution des phénomènes de violences lors des manifestations nécessite des réponses juridiques innovantes à mettre en oeuvre dans les meilleurs délais. Aussi, dans un souci de pragmatisme et dans le but de répondre aux attentes légitimes de nos forces de l'ordre, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte adopté sans modification par notre commission des lois.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un point au moins nous rassemble, à savoir la volonté de consolider le droit de manifester en démocratie.

Par quoi le droit de manifester, que ce pays pratique depuis deux siècles, est-il fragilisé ? Simplement, mais durablement depuis plusieurs années, par l'intervention de groupes organisés de combat urbain, qui entreprennent, à l'occasion de manifestations où ils s'engagent et contre l'avis de leurs organisateurs, des destructions systématiques et des agressions contre les policiers et les gendarmes. groupes, nous le savons, assurent leur dissimulation et leur anonymat, ce qui rend particulièrement difficile la répression pénale de leurs délits ; ils peuvent ainsi reproduire aussi souvent que possible ces méfaits. Le résultat qu'ils obtiennent fait déjà partie de nos habitudes de pensée et de débat. À l'issue d'une manifestation, le débat depuis plusieurs années sur le nombre de blessés et l'importance des dégâts, alors que l'appel à l'opinion démocratique que visait la manifestation se trouve détourné ou détruit. il faudrait analyser de façon un peu plus fine ce que sont ces groupes, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils propagent comme pensées.

que ces groupes organisés sont là pour défendre les droits de la personne et les principes de la République ; ils sont en action pour les combattre et les affaiblir. Il nous semble donc, conformément à la position d'une majorité au Sénat, puis d'une majorité à l'Assemblée nationale, qu'il convient d'ajouter des outils, des outils préventifs, à la protection du droit de manifester.

! Les rapports de police tout à fait circonstanciés expliquent que, si l'on avait voulu l'intercepter en pleine action, on aurait provoqué des scènes d'émeutes avec des dizaines de blessés. blessés. C'est là le descriptif exact de la façon d'agir de ces groupes, qui se sont méthodiquement préparés. Aussi, je crois vraiment que la sanction individuelle au travers de l'acte judiciaire est, hélas ! assez peu adaptée à ces situations.

vise d'abord à vérifier que ne s'approchent pas du lieu de manifestation des personnes équipées d'armes par destination. Est-ce favorable ou défavorable au droit de manifester ?

-dans des phases violentes de manifestation. C'est là une réponse à notre collègue Loïc Hervé, qui connaît bien la manière de travailler de la justice administrative.

L'interdiction individuelle de manifester qui sera prononcée par l'autorité administrative sur des données objectives pourra être contrôlée quasi instantanément par un juge. Cet outil juge. Cet outil de prévention à l'égard des personnes qui se sont organisées pour venir perturber de façon violente des manifestations est donc adapté. La mesure d'application de l'inscription dans le fichier des personnes recherchées est évidemment appropriée. Nous ajoutons, il est vrai, une sanction pénale supplémentaire, qui, elle, sera prononcée par le juge dans le cas de dissimulation volontaire du visage sur un lieu de manifestation. Ce texte, je l'ai souligné, donnera lieu à une évaluation par le Parlement.

de la V République que d'avoir prévu un contrôle volontaire de constitutionnalité actionné par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le Président de la République. Si ces quatre autorités de l'État ont reçu, depuis 1958, le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel, ce n'est pas prioritairement pour entraver l'application de la loi nouvelle ; c'est pour obtenir, avant

il me semble que- tous les commentaires sont naturellement les bienvenus, et leur pertinence sera d'autant plus aisée à apprécier d'ici à un mois environ, lorsque nous aurons la réponse finale -nous faisons là une application parfaitement orthodoxe des principes de nos institutions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a quelques mois, le président Macron arguait : « La démocratie, ce n'est pas la rue. Au contraire, c'est aussi cela la démocratie. En quoi cette proposition de loi répond-elle aux violences commises par certains individus dans les manifestations ? Les casseurs qu'elle prétend viser ne sont pas inquiétés outre mesure ces derniers temps, me semble-t-il, alors même que les forces de l'ordre ont les moyens de les arrêter en amont, avant qu'ils ne perpètrent leurs actes de violence et leurs dégradations. Épuisée par des mois de conflits sociaux, notre société est aujourd'hui scindée, morcelée. Par son refus de répondre aux revendications de nombre de Françaises et Français, l'exécutif a brisé la paix sociale. Là est le problème que vous ne voulez pas voir. Quelle ironie que ce texte du sénateur Retailleau, pour lequel le Gouvernement avait demandé un avis de sagesse au Sénat, Sénat, se soit tout à coup transformé, à son arrivée à l'Assemblée nationale, à la faveur du mouvement des « gilets jaunes », en un texte essentiel pour vous, monsieur le ministre droite sénatoriale et majorité présidentielle à l'Assemblée nationale vont adopter un texte conforme, faisant ainsi fi des grandes institutions internationales, qui ont récemment dénoncé l'escalade des violences anti-manifestants dans notre pays. ne se fera pas sans la grogne d'une cinquantaine de députés LaREM. Les articles 2 et 4 sont particulièrement préoccupants et ne respectent pas les obligations internationales de la France en matière de droits humains. L'article 2 instaure la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester à des personnes, sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire, avec une possible obligation de pointage et d'interdiction de se rendre à certains endroits. Dès lors, c'est à l'autorité préfectorale de justifier quelles « personnes constitueraient des menaces à l'ordre public ». Permettez-moi de douter du caractère objectif des éléments risquant de motiver la décision du préfet. Quels seront réellement les critères utilisés pour cibler tel individu et quels seront les signes distinctifs qui viendront fonder les suspicions de l'administration ? J'ai bien peur que des éléments simplistes tels que l'appartenance ethnique ou politique ne soient retenus et n'ouvrent pleinement la voie à l'arbitraire. L'article 4 instaure l'interdiction de se voiler le visage lors des rassemblements, sur la base de présomptions de troubles à l'ordre public. Doit-on rappeler ici que les gaz lacrymogènes se répandent dans l'air et ne touchent pas seulement leurs cibles désignées ? Doit-on condamner les passants et manifestants non violents qui auraient eu l'audace de se protéger les voies respiratoires par un masque ou un tissu, afin de ne pas inhaler de substances toxiques

Se donnant en apparence pour ambition de lutter contre la présence des casseurs dans les cortèges, cette proposition de loi cible finalement plutôt des personnes non violentes, à l'instar de ces nombreux « gilets jaunes », ... Non ! ... blessés et mutilés, mais aussi de notre collègue député

et que ce texte ne viendra en rien l'améliorer. Ce sont nos méthodes qu'il faudrait adapter aux réalités du terrain. faut jamais oublier que des textes de ce genre pourront être utilisés plus tard par des exécutifs totalement antidémocratiques et se transformer en simple interdiction de manifester. En préférant vous en remettre aux décisions administratives plutôt qu'aux instances judiciaires, c'est l'État de droit que vous mettez en péril. En décrétant des interdictions de manifester sur la base de « présomptions » particulièrement floues, c'est l'égalité des citoyens devant la loi que vous bafouez. Par l'instauration de responsabilité pénale et civile collective pour la dégradation de biens publics, c'est le principe d'individualité des peines qui est mis à mal. Souvenons-nous que nos acquis sociaux et nos libertés fondamentales sont nés dans la rue. Et c'est dans la rue qu'ils continueront à être défendus Au nom de l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui garantit symboliquement le droit de manifester, et au nom de la défense de l'État de droit, le groupe CRCE s'opposera résolument et en toute conscience à l'adoption de cette

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, le débat d'aujourd'hui ne peut pas, ne doit pas être escamoté. Certains souhaiteraient que nous ne parlions de cette proposition de loi que sous l'angle de la nécessaire sécurité sécurité des biens et des personnes. Pour ma part, je me refuse, au nom de mon groupe, à aborder ce texte uniquement sous ce prisme sécuritaire. Ce débat est plus important encore, car il s'agit d'un débat de valeurs et de principes républicains, et non pas seulement d'un débat pénal et juridique. Le contexte, d'abord. Notre pays a connu ces derniers mois une série de manifestations d'un nouveau type, chacun le reconnaît : non déclarées, souvent spontanées, souvent alimentées par le bouche à oreille moderne que sont les réseaux sociaux. seulement la question de la sécurité de ces manifestations a été posée à juste titre, mais aussi celle de la sécurité qui entoure ces manifestations. De nombreux et inacceptables débordements ont eu lieu malgré le dévouement dans l'action des forces de l'ordre, que je veux, à mon tour, saluer. Voilà le constat. Mais quelles conséquences politiques devons-nous en tirer face aux dégradations et aux blessés si nombreux dans ces manifestations, dans les deux camps d'ailleurs ? Faut-il conclure, comme nous le suggère la proposition de loi Retailleau-Macron, que la cause de ces violences se situerait d'abord dans l'exercice de ces manifestations ? Ou pouvons-nous avoir un peu plus de recul, en remarquant que la doctrine du maintien de l'ordre en France n'est peut-être plus adaptée à ce type de manifestations ? de loi, modifiée, comme nous le savons, par l'Assemblée nationale, est un texte de circonstance, qui n'apporte pas de solutions réfléchies, conformément à ce que devrait être l'objectif de toute loi. Par ailleurs, le recours prévu du Président de la République devant le Conseil constitutionnel constitue, selon moi, mais aussi, me semble-t-il, pour beaucoup d'entre nous, une intrusion anormale, j'y insiste, dans le débat parlementaire.

La liberté de manifester découle de la Constitution et aussi de l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit la libre communication des pensées et des opinions.

sans faille. Nous sommes évidemment favorables à ce que les violences ayant lieu au cours des manifestations soient évitées et que, lorsqu'elles ont lieu, leurs auteurs soient poursuivis et condamnés, car ce n'est qu'ainsi que la liberté de manifester peut être pleinement garantie. Toutefois, cela ne peut se faire dans le respect des règles et principes constitutionnels, des droits et libertés que la Constitution garantit. Et c'est bien une remise en cause du droit de manifester qui nous est proposée dans l'article 2 de cette proposition de loi. Avec votre texte, monsieur Retailleau, monsieur Castaner, et sans revenir davantage sur les autres articles que nous contestons, comme l'a rappelé très justement notre collègue Jérôme Durain, vous créez un nouveau pouvoir administratif, extensif, dont nous pouvons redouter l'arbitraire, puisqu'il vise à interdire à certaines personnes de manifester, et donc de s'exprimer. Cette loi d'arbitraire suspecte de fait le manifestant d'être manifestant pour casser. Cette loi d'arbitraire assimile les notions de manifestants et de délinquants menaçant l'ordre public. Mais au nom de quoi, mes chers collègues ? Au nom de la sécurité ?

Il existe enfin tout ce qui est utile pour organiser des manifestations dans de bonnes conditions, lorsque l'on ne méprise pas et ne rabaisse pas sans cesse, bien sûr, les corps intermédiaires. Nous voulons réaffirmer ici que le droit de manifester s'inscrit dans le prolongement de la liberté d'expression, si fondamentale à notre République. Prenons un exemple. Pourrions-nous accepter, mes chers collègues, qu'une personne, bien qu'elle ait pu abuser de sa liberté d'expression par des propos diffamants ou d'autres délits,

qui ne serait qu'un pouvoir arbitraire, monsieur Grosdidier, supprimant ainsi la liberté d'expression de certaines personnes. Votre proposition de loi fragilise le droit de manifester, que vous le vouliez ou non. Dans l'histoire de notre pays, ce droit a été complexe à obtenir, chaotique, difficile à s'écrire totalement. Ce droit de manifester a longtemps été inachevé, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel reconnaisse enfin cette liberté. Remettre aujourd'hui en cause cette liberté, mes chers collègues, c'est revenir au temps de la République inaboutie, celle qui ne reconnaissait pas le droit de manifester comme un prolongement du droit d'expression. Remettre en cause le droit de manifester, comme vous le faites aujourd'hui, c'est affaiblir encore un peu plus le discours de la France sur les droits de l'homme, déjà mis à mal, puisque nous subissons, comme l'a indiqué Mme Benbassa, des enquêtes du Conseil de l'Europe et de l'ONU sur la gestion des manifestations qui émaillent notre pays. chers collègues, il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts dans des manifestations, comme c'est le cas dans certains États autoritaires, pour s'inquiéter de la privation des libertés et du danger pour la démocratie que représentent les interdictions générales. C'est pour défendre la liberté que, dès l'origine, nous avons combattu ce texte. Nous l'avons combattu, dans sa version initiale, à l'automne, ici même au sein de la Haute Assemblée. Nous le combattons dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, alors que la majorité des députés et le Gouvernement ont joué avec le feu et sont en train de se brûler. Nous le combattrons, à sa sortie du Sénat, si nous n'arrivons malheureusement pas à vous convaincre. Nous le combattrons jusqu'au bout, tant qu'il en existera un morceau dans notre droit, si jamais ce texte devait être promulgué en l'état. Très bien ! Il existe des principes républicains dans notre pays, nous l'espérons encore du moins. Que la justice, celle qui est rendue au nom du peuple, soit la seule à pouvoir décider d'entraves durables aux libertés est, pour nous, un principe essentiel, un principe intangible Et toujours- toujours ! -, mes chers collègues, vous nous trouverez pour nous élever contre des lois d'arbitraire qui entravent les citoyens. Un citoyen ne peut être pleinement citoyen que s'il peut jouir pleinement de ses droits et libertés. L'État ne peut pas décider seul de qui serait ou non pleinement citoyen. Aussi, et j'en viens à ma conclusion, je vous invite, avant d'émettre votre vote sur ce texte, à écouter et entendre cette phrase qui résonne comme une alerte : « Le droit et la loi, telles sont les deux forces :

de leur antagonisme naissent les catastrophes. » Mes chers collègues, merci à Victor Hugo de nous tracer encore une fois le chemin

La séance est reprise.

et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, depuis le 22 février dernier, une grande partie du peuple algérien est descendue dans la rue pour s'opposer à un cinquième mandat du Président Bouteflika- dans un esprit pacifique, il faut le souligner. Cette mobilisation, inédite sous cette forme depuis très longtemps, a évidemment contribué à faire évoluer les positions du pouvoir, d'abord lorsque le Président Bouteflika a annoncé qu'il ne terminerait pas son cinquième mandat s'il venait à être réélu, puis, hier soir, lorsqu'il a annoncé renoncer à une nouvelle candidature, invoquant cette fois son âge et sa santé. Si cette annonce satisfait à court terme les revendications des manifestants pour une modernisation du système politique, elle ne répond pas aux attentes fondamentales du peuple algérien, ne soyons pas naïfs ! Aujourd'hui, la contestation pourrait évoluer vers une volonté de changement plus large. Le scrutin présidentiel devrait avoir lieu après une conférence nationale « inclusive et indépendante », représentative de toutes les composantes de la société, avec, pour mission, d'élaborer avant la fin de l'année un projet de Constitution à soumettre au référendum. Cela revient à reporter l'élection présidentielle à une date non fixée. Le Président Emmanuel Macron a accueilli avec satisfaction ces annonces, appelant au passage « une transition d'une durée raisonnable ». Or, on le sait, nos deux pays entretiennent depuis longtemps des relations complexes, passionnelles, mais étroites. Pourriez-vous, monsieur le Premier ministre, nous préciser la position de votre gouvernement après ces dernières évolutions ?

que l'on peut qualifier les relations entre la France et l'Algérie, parce que notre histoire est, à bien des égards, une histoire commune, parce qu'elle a connu des moments de lumière et des moments d'ombre, parce que

Je veux le dire, même si personne n'a de doute sur le sujet, l'Algérie est un État souverain, et nous respectons totalement cette souveraineté. Les évolutions récentes de la situation

Le Président Bouteflika a fait savoir hier, dans son message à la nation, qu'il renonçait à se présenter à l'élection présidentielle initialement prévue le 18 avril. Il a proposé les jalons d'une rénovation du système politique algérien, avec un remaniement ministériel, qui s'est traduit par la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un vice-Premier ministre, l'organisation d'une conférence nationale, dont les travaux doivent se conclure d'ici à la fin de l'année et devraient déboucher sur l'adoption, par référendum, d'une nouvelle Constitution, et enfin- après tout cela -la tenue de l'élection présidentielle à laquelle lui-même ne serait pas candidat. Nous avons salué ces Nous avons salué ces derniers développements. Ces annonces interviennent à l'issue de plusieurs semaines de manifestations à travers tout le pays, qui ont vu des millions d'Algériens et d'Algériennes exprimer, dans le calme, dans la dignité, leurs aspirations. Nous notons aussi que ce civisme des manifestants s'est accompagné d'une grande retenue des forces de l'ordre, lesquelles ont été exemplaires. Nous souhaitons que cet esprit de responsabilité, relevé par l'ensemble de la communauté internationale, puisse perdurer afin que se mettent en place les conditions d'une solution démocratique. Ce qui doit maintenant s'engager, c'est une dynamique à même de répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, avec, surtout, l'élaboration d'un calendrier politique de transition raisonnable,

tant vos arguments peinent à convaincre ! Le privé serait, selon vous, meilleur gestionnaire que le public. Faux ! ADP est le deuxième groupe aéroportuaire d'Europe, en passe de devenir le premier, selon de nombreuses études. L'État n'aurait pas vocation à entrer dans le jeu concurrentiel. Pourtant, vous proposez de privatiser un service public national, doublé d'un monopole naturel. Il faut 250 millions d'euros pour financer le Fonds pour l'innovation. Or les sociétés ADP, Engie et la Française des jeux, toutes privatisées par la loi Pacte, représentent plus de 700 millions d'euros de dividendes. Et que dire des recettes qui pourraient être être attendues d'un rétablissement de l'ISF ! L'État gardera-t-il une part du capital d'ADP ? À la veille de la privatisation, rien n'est encore décidé ! Enfin, vous ne tirez pas la leçon de l'avis du rapporteur public de la cour administrative d'appel de Paris, qui préconise, après les critiques acerbes de la Cour des comptes, l'annulation de la privatisation, ô combien douteuse, de l'aéroport de Toulouse. Dès lors, loin de la théorie du complot, il s'agit de donner des réponses claires à la représentation nationale et à nos concitoyens, qui ne comprennent pas qu'on puisse les spolier, dans la durée, d'un bien d'intérêt national stratégique, financé par l'argent du peuple. La vérité doit être dite ! Vinci n'a pas eu Notre-Dame-des-Landes, mais recevra une part de la somme de 1 milliard d'euros qui sera versée aux actuels actionnaires minoritaires. Oui ou non, Vinci utilisera-t-il l'argent public pour acheter les biens du peuple ?

Elle structure de plus en plus les débats politiques, en pour ou en contre ; elle structure aussi les relations internationales- notre pays a donné l'exemple, je le rappelle, avec la signature de l'accord de Paris, voilà plus de trois ans.

En février, déjà, de nombreux lycéens et étudiants de notre pays ont rejoint ce mouvement de grève en faveur du climat. Ce vendredi, selon toute vraisemblance, le mouvement devrait s'amplifier, avant de nouvelles marches pour le climat prévues le week-end prochain. Ce mouvement de la jeunesse, spontané et international, doit faire réagir les pouvoirs publics. Il est temps de comprendre, non seulement l'inquiétude de ces jeunes, mais aussi leur aspiration à un changement global clair. Il faut un engagement fort de notre société face à cet élan de la jeunesse, aussi généreux que lucide. noté, monsieur le Premier ministre, que l'éducation nationale organiserait des débats dans les lycées pour faire remonter les idées des lycéens sur le sujet.

ou, du moins, contenir le réchauffement climatique, qui, loin d'un fantasme de professeur Cosinus, est bien une réalité ? Quelles mesures allez-vous prendre pour que la France respecte ses engagements de 2015 ? Enfin,

J'étais ce matin à Tours, pour discuter, dans le cadre du grand débat, avec des jeunes d'une école de la deuxième chance. Lorsque l'on assiste pendant un temps long à de tels échanges, on voit bien que chacun a des idées pour le quotidien, idées qu'il faut structurer pour le futur.

grâce à la mobilisation des citoyens et du Gouvernement. Ce qui va se passer vendredi aura beaucoup d'importance. Sachez que, le 5 avril prochain, nous réunirons l'ensemble des représentants lycéens de France pour, précisément, structurer les propositions émanant de la jeunesse.

groupe Les Indépendants - République et Territoires. Ma question porte sur l'accompagnement des entreprises qui subissent la crise du diesel. En sept ans, la part du diesel est passée en France de 73 % à 35 %. Les sous-traitants souffrent, notamment ceux de Renault. 15 000 emplois, sur les 38 000 de la filière, qui sont menacés. En juillet 2018, j'ai interrogé M. Le Maire. Il s'est engagé à accompagner les industries pour défendre les emplois, dont les Fonderies du Poitou, implantées à Châtellerault. a annoncé que le fonds d'aide industrielle, doté de 10 milliards d'euros, financerait la diversification de ces entreprises. Le 16 octobre à l'Assemblée nationale, il s'est une nouvelle fois engagé à accompagner la transformation des Fonderies

L'État est actionnaire, est-ce le seul engagement obtenu ? L'offre de reprise, qui a votre soutien, prévoit de ne conserver qu'un emploi sur deux, tout en faisant appel à des intérimaires pour honorer les commandes. Ce n'est pas sérieux ! Hier, vous avez réuni les constructeurs, équipementiers, syndicats, et des présidents de région. Belle initiative ! Mais il faut que cela débouche sur des mesures concrètes. Après un an de crise, pouvez-vous rassurer les 850 salariés ? L'État continuera-t-il à faire pression sur Renault ? Allez-vous utiliser les fonds d'aide industrielle pour consolider les offres de reprise de ces deux sites ? Allez-vous réhabiliter le diesel « propre », moins polluant aujourd'hui que l'essence ?

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. L'annonce d'une baisse drastique du budget de la politique agricole commune, la PAC, a suscité une onde de choc. Elle se traduira par une perte d'environ 8 milliards d'euros pour l'agriculture française, et pas seulement à cause du Brexit. Quels revenus pour nos agriculteurs demain ? Plus grave encore, dans le nouveau modèle imaginé par la Commission européenne, ce sont désormais les États qui définiront en grande partie les conditions à respecter pour bénéficier des aides agricoles. C'est donc le risque d'une renationalisation de la PAC, c'est-à-dire d'un retour à vingt-sept politiques agricoles nationales différentes. Un tel scénario signifierait toujours plus de concurrence avec nos voisins, toujours plus de contrôles de la Commission européenne, toujours plus de complexité ! Le 14 février dernier, les commissions des affaires européennes et économiques du Sénat ont ont adopté, à l'unanimité, une nouvelle proposition de résolution européenne sur la PAC. Monsieur le ministre, allez-vous saisir cette ultime opportunité pour remettre à plat cette réforme de la PAC, mal engagée ? Aucun Président de la République, aucun des ministres qui vous ont précédé n'ont cédé sur le sujet. Alors que l'Inde, la Chine ou les États-Unis n'hésitent pas à mettre un « pognon de dingue » dans leur agriculture, ne laissez pas l'histoire se souvenir de vous comme le ministre qui aura fait renoncer la France et l'Europe à leur ambition agricole !

Seuls les dossiers agréés avant cette date bénéficieront d'un financement. Cela, à cause de plusieurs erreurs qui auraient pu être évitées avec un minimum de préparation ! La refonte du système de recouvrement de la contribution à la formation professionnelle a entraîné un assèchement de la collecte, qui est passé de 72 millions d'euros l'an passé à 40 millions d'euros cette année. Cette situation s'impose, de façon brutale, à tous les organismes de formation professionnelle concernés, qui se trouvent dans une position critique, étranglés. Nous sommes nombreux à avoir été saisis de ce scandale par les chambres de métiers et de l'artisanat, les syndicats professionnels, les organismes de formation ... Autant d'organisations professionnelles qui expriment une très grande inquiétude. La formation professionnelle est essentielle à nos entreprises artisanales. On ne peut imaginer qu'elle soit suspendue jusqu'à une date indéterminée, mettant par la même occasion de nombreux emplois en péril.

des finances publiques, en application de la loi Travail. Cette modification des modalités techniques de collecte a entraîné des difficultés de trésorerie pour le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale, ainsi que pour les conseils en formation. En effet, l'ordre national des experts-comptables a eu une interprétation de cette modification qui a conduit les artisans à ne pas payer l'intégralité de la cotisation dont ils étaient redevables.

dans la loi, les chefs d'entreprise en question sont bien redevables de ces cotisations. Après, on peut essayer de trouver une solution politique visant à pondérer ces cotisations, qui sont effectivement

de la santé. C'est un fait : la question de la pauvreté en France est très préoccupante, et ce depuis de très nombreuses années. On compte près de 9 millions de personnes vivant en situation de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Ce sont autant de situations d'exclusion et de difficultés d'insertion. La délégation interministérielle à laquelle j'ai participé a rendu ses conclusions : il est temps de traduire dans les faits le plan Pauvreté, qui allie « prévention » et « accompagnement ». C'est dans ce cadre, madame la secrétaire d'État, que vous lancez les travaux sur le revenu universel d'activité. L'objectif est d'améliorer la protection sociale, de lutter contre les non-recours, notamment en simplifiant les démarches et en proposant une refonte de certains minima sociaux, tels que le RSA, la prime d'activité, voire les aides au logement. Il faudra s'interroger sur l'ensemble des personnes précaires, les étudiants, les retraités, et je n'oublie pas le monde agricole. Ces travaux s'appuieront, à n'en pas douter, sur les points de vue des acteurs concernés, tels que les CAF, les collectivités territoriales, les associations de solidarité,

fusionnant le plus grand nombre possible de prestations. Comme vous venez de l'expliquer, ce projet nécessite une expertise très importante. C'est pourquoi je réunirai ce jeudi, aux côtés de Fabrice Lenglart nommé rapporteur général, le comité interadministratif destiné à lancer les travaux techniques. La réforme que je porte est essentielle. Elle doit permettre de mieux répondre à cinq impératifs : l'impératif de dignité pour permettre à ceux qui n'ont pas ou peu de revenus professionnels d'être protégés de manière adéquate ; l'impératif de simplicité d'accès au droit pour lutter, comme vous l'avez dit, contre le non-recours droits ; l'impératif de transparence pour permettre aux allocataires de prévoir l'évolution de leurs revenus et les inciter à reprendre une activité ; l'impératif d'équité pour garantir une égalité de traitement aux personnes se trouvant dans des situations équivalentes ; enfin, l'impératif de responsabilité autour d'un contrat d'engagement réciproque rénové entre l'État et les bénéficiaires pour que chacun soit accompagné vers une activité. Cette réforme sera d'une grande ampleur. Il est donc indispensable de mener un travail collectif de concertation et d'analyse pour définir précisément les contours et les paramètres de cette future prestation. les différents scénarios, de façon à ce qu'aucun choix ne soit préempté. De nombreuses prestations sont potentiellement concernées : le RSA, l'APL, la prime d'activité, mais aussi le minimum vieillesse, l'AAH ou l'ASS. Nous devrons aussi nous poser la question des jeunes et de l'intégration des 18-25 ans dans ce dispositif. Au-delà de ces Au-delà de ces travaux techniques, une concertation institutionnelle et citoyenne sera lancée à partir du printemps, et pour toute l'année 2019. J'ai demandé à ce que cette concertation associe toutes les parties prenantes- vous en avez cité quelques-unes - : les collectivités, les CAF, les MSA, les associations, mais aussi nos concitoyens. Aussi, j'invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à participer à cette concertation pour élaborer un texte qui sera présenté en 2020. La parole

l'échec de la négociation sur la réforme de l'assurance chômage était annoncé. Née de la volonté du chef de l'État, supplantant celle du Gouvernement, annoncée devant le Congrès de Versailles, concrétisée par le dépôt d'un amendement tardif lors de l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel par le Sénat, la renégociation anticipée de la convention d'assurance chômage, alors que la précédente ne datait que du mois de juillet 2018, n'était pas placée sous les meilleurs auspices. Déjà, le sentiment que le Gouvernement ne respectait pas le débat démocratique, non

que de leur demander de négocier sur un bonus-malus d'ores et déjà acté par le Président de la République. Ma question est la suivante : en supprimant les cotisations chômage des salariés pour les remplacer par de la CSG, évoluant d'une logique d'assurance à une logique de solidarité, n'avez-vous pas implicitement prémédité la déresponsabilisation des syndicats et tronqué une négociation à laquelle vous n'avez vous-même peut-être jamais cru, signant ainsi la quasi-fin du paritarisme dans notre pays ?

le Gouvernement a fait le choix de placer le travail au coeur du projet politique que nous défendons. Lequel ? Vous l'avez rappelé, nous avons demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir des négociations sur l'assurance chômage, qui n'ont malheureusement pas abouti.

deux objectifs : lutter contre la précarité et inciter au retour à l'emploi. L'enjeu est d'ailleurs double : d'abord, inciter les entreprises à proposer des contrats de travail plus longs et privilégier les embauches en CDI pour « déprécariser

ce que nous vivons est bien différent ! En fixant un tel cadre aux partenaires sociaux, c'était immanquablement la chronique d'une mort annoncée de la nouvelle négociation de l'assurance chômage ... Eh oui ! ... et, je le crains, la chronique d'une mort annoncée de cinquante ans de paritarisme dans notre pays. La parole est

d'une maladie chronique qui touche uniquement les femmes et qui se manifeste par des douleurs gynécologiques récurrentes et souvent handicapantes. Cette maladie reste encore trop méconnue aujourd'hui. Le diagnostic est réalisé avec un retard moyen de cinq ans, ce qui laisse la maladie gagner du terrain. Elle est encore trop souvent révélée après un bilan de fertilité, donc à un stade bien avancé, car c'est une maladie qui ne se guérit pas : 40 % des femmes atteintes sont infertiles. Les causes de la maladie ne sont pas réellement identifiées et les traitements disponibles ne sont pas pleinement satisfaisants. On peut facilement mesurer les souffrances physiques et morales de l'endométriose pour les femmes concernées et leur entourage. Certains témoignages de femmes font état de situations d'isolement et de détresse, allant même jusqu'à compromettre leur vie professionnelle. Nous avons beaucoup à faire pour améliorer la qualité de la prévention de cette maladie ces prochaines années. Ce chantier est devant nous. Il faut ici saluer l'engagement décisif des associations, notamment EndoFrance, qui ont voulu briser le silence et médiatiser cette maladie de l'ombre, par définition, si intime, et donc, si sensible. ces associations se sont mobilisées lors de la semaine européenne de l'endométriose, des campagnes de sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux. Le Gouvernement a présenté une feuille de route ambitieuse le vendredi 8 mars pour faire de l'endométriose une priorité de notre politique de santé publique, davantage qu'un simple drame privé. Pourriez-vous indiquer quelles en sont les principales avancées, nous communiquer, si cela est possible, des éléments de calendrier et la manière dont les élus y seront associés ? La parole

et trop silencieuse. Elle est encore trop méconnue des femmes, mais aussi des professionnels, ce qui engendre souvent des retards de diagnostic, des errances médicales, dont les femmes sont les premières victimes. À l'occasion de la journée internationale des femmes et pour clore la semaine européenne de prévention et d'information consacrée à cette maladie, Agnès Buzyn a visité vendredi dernier le centre de l'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph et y a annoncé le lancement d'un plan d'action s'articulant autour de trois axes. Notre premier objectif est de détecter précocement cette maladie, en intégrant la recherche de signes d'endométriose lors de consultations dédiées à la santé sexuelle des jeunes femmes entre quinze et dix-huit ans et en renforçant la formation sur les signes d'alerte, le diagnostic et la prise en charge dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé concernés. Le deuxième axe vise à mieux accompagner les femmes et à rendre simples et cohérents les parcours de soins. Aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, les parcours de soins sont trop erratiques. La prise en charge de la douleur et des troubles de la fertilité devront aussi faire l'objet d'une vigilance particulière, afin de mieux répondre aux légitimes inquiétudes. Enfin, nous voulons mieux informer sur cette maladie encore trop méconnue. En complément des campagnes de communication et des associations, il nous faut mieux faire connaître la maladie et sa prise en charge, en mobilisant notamment le service sanitaire des étudiants en santé, pour informer les élèves dans les collèges et les lycées sur la maladie et sensibiliser les futurs professionnels de santé. L'ensemble des parties prenantes sera associé aux travaux de mise en place de ce plan d'action. Notre objectif est donc simple : apporter des réponses concrètes aux femmes touchées par cette maladie complexe et douloureuse, qui la vivent aujourd'hui souvent en silence, faute de diagnostic ou de prise en charge adaptée.

1,4 million d'entreprises artisanales. Nous sommes tous fiers de nos artisans, de leurs compétences, de leur savoir-faire et de leur professionnalisme. Ce sont eux qui créent les richesses, qui créent l'emploi, qui accompagnent les jeunes, qui assurent la formation des entreprises.

un déficit de plus de 30 millions d'euros, parce que 177 000 adresses d'entreprises ont mystérieusement disparu des fichiers. Cela n'est pas

Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la garde des sceaux, au terme du grand débat voulu par M. le Président de la République pour répondre à la crise des « gilets jaunes il ne vous aura pas échappé que, pour une grande majorité d'entre eux, nos concitoyens doutent de la capacité des seules institutions à apporter des réponses aux grandes questions du moment. Au-delà du doute, nous pouvons considérer qu'il y a même, dans leur expression, une forme de défiance à l'égard de la communication des institutions publiques comme de celle des grandes entreprises privées, faisant leur la phrase devenue célèbre d'une humoriste : « On ne nous dit pas tout ! C'est pour répondre à ce besoin d'une information objective que des femmes et des hommes se sont exposés pour rendre publics des faits répréhensibles par notre droit. Les plus connus, Alain Robert, Hervé Falciani, Stéphanie Gibaud ou encore Irène Frachon, peuvent être considérés comme les précurseurs de ceux qu'on appelle communément les « lanceurs d'alerte Dans ces conditions, l'accord trilogue- Parlement européen-Conseil-Commission européenne -intervenu hier, 11 mars, sur la directive relative aux lanceurs d'alerte, sur le fondement de la proposition de notre collègue eurodéputée Virginie Rozière, doit être salué.

La France a toujours soutenu le principe d'un texte unique, au champ d'application large, couvrant de très nombreux domaines d'action de l'Union, y compris, d'ailleurs, la fiscalité. Aujourd'hui, l'essentiel de la directive fait donc l'objet d'un accord avec le Parlement européen. Il restait un point de divergence sur la hiérarchie des canaux de signalement. Oui ! Le Conseil, au sein duquel la position de la France n'était d'ailleurs pas isolée, souhaitait conserver comme principe-

tenu à une obligation de stricte confidentialité. Nous pensons en effet que c'est ainsi que l'on peut mettre un terme le plus rapidement possible à une violation dénoncée. C'est d'ailleurs le cas dans la majorité des situations. Ce principe était assorti d'exceptions extrêmement larges,

la France ne souhaite pas retarder l'adoption de ce texte. C'est pourquoi nous avons accepté de supprimer cette hiérarchie des canaux de signalement. Nous allons ainsi parvenir à un texte assurant une protection maximale des lanceurs d'alerte, tout en instituant un mécanisme solide juridiquement et proportionné aux différents niveaux de gravité des signalements effectués. Nous touchons au but avec un accord en vue d'ici à vendredi

depuis lesquelles je m'exprime et nombre de parlementaires se reconnaissent difficilement dans les arguments que vous aviez alors avancés pour justifier votre timidité sur le sujet. Nous nous reconnaissons davantage dans cette citation de Jean Jaurès : « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire

Difficultés économiques et sociales, disparition progressive des services publics dans les communes, poids de la fiscalité, sentiment d'injustice devant les inégalités sociales : les motifs de préoccupation sont nombreux et alimentent parfois la colère des Français. Comme vous, mes chers collègues, je sens depuis longtemps monter le souffle de la contestation dans mon département de Loir-et-Cher, et ce aussi bien au sein de la population que chez les élus locaux. L'une des origines de ce malaise se trouve dans la fracture territoriale, qui ne cesse de se creuser entre la France des grandes villes et celle des campagnes et des petites villes. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité du quotidien. Dans les petites communes rurales, les habitants voient leurs services publics disparaître et les distances de trajet s'allonger. Le sentiment d'isolement, et même d'abandon, gagne nos campagnes. Ce sentiment est partagé par nos élus locaux, extrêmement sollicités, mais qui manquent cruellement de moyens et de soutien. En ces temps difficiles où les principes fondateurs de notre République sont remis en question, c'est précisément le moment de nous appuyer sur le formidable tissu d'élus locaux pour rétablir l'équilibre territorial. Pour ce faire, il est primordial de réaffirmer et de renforcer le principe de décentralisation inscrit à l'article premier de notre Constitution.

Aussi, ma question est simple : ferez-vous de la décentralisation la clé de voûte de la révision constitutionnelle à venir ? La parole

et reconnaissons que l'oeuvre collective mise en oeuvre depuis quelques années n'a pas tout à fait abouti, ils souhaitent davantage de lisibilité. L'enchevêtrement d'un certain nombre de compétences, la succession d'un certain nombre de réformes n'ont pas clarifié les choses. Les citoyens ont besoin de lisibilité, parce qu'ils ont besoin de pouvoir identifier les responsabilités. Il n'y a pas de lisibilité possible sans identification des responsables,

je voudrais saluer la présence dans notre hémicycle, pour sa première séance de questions au gouvernement, de Mme Marie-Pierre Richer, devenue sénatrice du Cher en remplacement

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.

sans vouloir prêter d'intentions cachées à ses auteurs, il est vraisemblable que le mouvement des « gilets jaunes » a empêché cette proposition de loi de disparaître dans les limbes de la navette parlementaire.

Nous considérons comme vous, mes chers collègues, que le maintien de l'ordre garantit l'exercice pacifique du droit de manifester. Que les violences qui agitent certains cortèges jettent le discrédit sur l'ensemble des manifestants, tandis que d'autres foules, de l'autre côté de la Méditerranée font preuve Maintenant que cette proposition de loi est devenue un des véhicules législatifs visant à apporter une réponse à la crise des « gilets jaunes », il nous faut composer avec cette ruse de l'histoire qui transforme parfois les textes de circonstance en lettres de loi. Sur l'encadrement des manifestations, les questions sont pourtant nombreuses et mériteraient que l'on y consacre plus de temps. Faut-il, par exemple, revoir la procédure de déclaration en préfecture, dès lors qu'elle n'est pas toujours respectée, la définition de l'attroupement ? Une zone grise de la manifestation non déclarée, située entre la manifestation déclarée et l'attroupement, s'est développée dans la pratique, faute d'une base légale suffisante pour s'y opposer. Voilà un problème auquel il faudrait aussi Si l'on s'en tient aux seules dispositions que comporte ce texte, d'importantes questions de constitutionnalité et d'applicabilité restent encore en suspens, comme vous l'avez courageusement souligné, madame la rapporteure.

Je le répète, nous sommes nombreux ici à vouloir apporter des réponses utiles aux problèmes de violence que vous pointez, mais pas de cette façon, et pas maintenant. Mes chers collègues, je crois important de redire que chaque fois que le Parlement se dessaisit de sa compétence, il porte atteinte à son utilité, au moment où certains voudraient la mettre en question. Le Sénat, en particulier, s'est toujours honoré à se poser en « gardien des libertés », comme le disait notre ancien collègue François Pillet avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, rassemblons-nous autour de ce dessein, pour faire honneur à notre fonction de législateur de plein exercice. Montrons, par notre débat, que le bicamérisme est essentiel à notre démocratie parlementaire, plutôt que de nous en remettre fébrilement à l'examen du juge constitutionnel. constitutionnel l'expose lui-même dans un considérant de principe qu'il a posé depuis longtemps, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur. Autrement dit, il nous faut revenir à l'« acte de légiférer », comme le disait notre collègue Philippe Bonnecarrère en commission des lois, la semaine dernière. À l'Assemblée nationale, certains de nos collègues députés ont d'ailleurs exprimé leur volonté de parvenir à une rédaction plus proche de celle que nous avions adoptée en première lecture. Monsieur le ministre, le Gouvernement lui-même avait également alors reconnu le caractère inachevé de ce texte. Comme l'indique l'objet du sous-amendement n° 248, n° 248, « compte tenu de la date de dépôt de cet amendement, des améliorations pourront être apportées à la rédaction de ces dispositions dans le cadre de la navette parlementaire ». Il revient à présent à chacun d'entre nous de voter en conscience, plutôt que de vouloir chercher à prémunir l'autre assemblée contre ses états d'âme.

Nous espérons que cela permettra de répondre à nos principales préoccupations, qui portent sur l'effectivité du recours contre les interdictions administratives de manifester, et que des modifications permettront de se prémunir contre d'éventuels dévoiements de ces nouveaux dispositifs. Nous avons d'ailleurs déposé plusieurs amendements en ce sens. Les Français demandent légitimement à retrouver la paix civile.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues,

qu'il faut que nous saisissions cette occasion, par souci d'efficacité, par esprit de responsabilité, pour donner à nos forces de l'ordre, à la République, à la démocratie, les moyens de se protéger. J'ai entendu Patrick Patrick Kanner, président du groupe socialiste et républicain, faire appel à la grande figure tutélaire de Victor Hugo ; il me permettra d'y faire référence moi aussi. Hugo disait : « La République affirme le droit, mais elle exige le devoir. » De quel droit s'agit-il en

un dilemme : interdire les manifestations ou éradiquer ceux qui sont très violents et qui dévoient ce droit pour casser, pour piller, pour blesser, pour propager une haine « anti-flics » qui n'est autre que la haine de la République, de la démocratie.

que nous prenions les mesures législatives nécessaires. Encore une fois, on ne peut pas laisser ces minorités détourner ce qui est un droit d'expression pour le retourner contre l'État de droit. Ce grand retournement, ce retournement délétère,

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, il y a quelques mois, lorsque le Sénat examinait cette proposition de loi, nous étions loin de nous douter que l'actualité allait lui donner de l'importance. Nous n'étions guidés par un simple impératif : mettre fin à l'impunité chronique des casseurs. Le Sénat n'avait pas fait que réagir à chaud : il avait anticipé les problèmes qui gangrènent notre société en proposant des solutions pratiques. Je veux saluer ici l'initiative de Bruno Retailleau : si ce texte avait été adopté à temps, dès après sa transmission à l'Assemblée nationale, certains problèmes auraient pu être évités. regard du débat sur les institutions, nous avons là un exemple de l'utilité du Sénat. À bon entendeur ... Sous l'effet des circonstances, il y a eu une conversion salutaire du Gouvernement Nous avons besoin de cette proposition de loi, » a clairement dit le ministre de l'intérieur, que je salue. En effet, il a fallu plusieurs samedis marqués par des violences pour que l'exécutif reconnaisse la nécessité d'un dispositif approprié, au point même de parler de « loi anti-casseurs »- je cite de nouveau le ministre. Oui, au-delà de la victoire du bon sens, c'est bien celle des mots que je voudrais saluer. Une sémantique trop prudente anesthésie les consciences et empêche toute action. Lutter contre des délinquants et des criminels, ce n'est pas empêcher les manifestations. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité des personnes et des biens : elle est la raison d'être des pouvoirs publics et de la politique. Ne risquons pas la vie des policiers, des manifestants, des commerçants, au nom de fausses pudeurs. Il est anormal de voir, à chaque manifestation, les casseurs échapper aux poursuites et aux sanctions. Il y a, hélas ! une impunité chronique des brutes et des voyous, qui ne comprennent qu'un seul langage : celui de la force. Mais que diable faut-il faire pour aller en prison dans ce pays ? Le jet de boules de pétanque et de cocktails Molotov est déjà un acte insurrectionnel. Les auteurs non plus des délinquants, mais des criminels. Osons les qualifier ainsi ! À Paris, nous ne pouvons plus supporter ces fins de manifestations où des commerçants ont été attaqués, leurs commerces saccagés et pillés, des monuments profanés. Des immeubles ont même été incendiés ! Les conséquences auraient pu être encore plus dramatiques. Je veux saluer tous mes collègues maires d'arrondissement, de tous bords, qui se sont heurtés à une gestion parfois inefficace de l'ordre public. Faut-il attendre le pire pour agir ? L'impunité des casseurs peut se transformer en permis de tuer si l'on persévère dans cette lâcheté L'article 2 permet aux préfets de prononcer des interdictions de manifester et, en cela, il ne fait qu'étendre une solution déjà appliquée dans les stades et qui a prouvé son efficacité. L'interdiction administrative remédie à la lenteur de la justice. Alors que les décisions judiciaires peuvent se faire attendre des années, le temps d'une réponse adaptée se mesure en jours. Les personnes interdites de manifestation doivent être recensées dans un fichier. L'Assemblée nationale a même proposé que ce traitement relève du fichier des personnes recherchées, le FPR. La création d'un délit de dissimulation du visage dans une manifestation est aussi une nécessité incontournable

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a vingt-huit ans, je rendais mon uniforme de la gendarmerie après avoir servi militairement notre pays pendant un quart de siècle. Aussi est-ce avec gravité et émotion que je prends la parole aujourd'hui. Depuis de nombreux mois, nos forces de sécurité sont victimes d'une nouvelle forme de violence. Des individus armés et parfaitement organisés s'infiltrent dans des manifestations pour en découdre. Ces délinquants sont là pour en découdre. Ces délinquants sont là pour blesser, mutiler nos policiers et nos gendarmes. Ils s'en prennent à nos institutions et n'hésitent pas non plus à piller et à dégrader les biens privés ou publics. privés ou publics. Les chiffres sont alarmants : depuis le début du mois de novembre 2018, 430 gendarmes et plus de 1 000 policiers ont été blessés, certains gravement, voire très gravement. Notre arsenal juridique n'est plus adapté à ce nouveau contexte de violence, et l'occasion nous est enfin donnée d'y remédier. Permettez-moi de saluer le travail du président Bruno Retailleau, qui est à l'initiative de cette loi dite « anti-casseurs d'une première lecture à l'Assemblée nationale, ce texte a été amendé. Nos collègues députés ont d'ailleurs conservé l'esprit du dispositif et n'ont pas totalement dénaturé les principales mesures de la proposition de loi. c'est bien là la preuve de l'utilité de notre institution, ainsi que de la nécessité d'un dialogue entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le message, je l'espère, sera entendu en haut lieu. Toutefois, le Président de la République a fait savoir qu'il saisirait le Conseil constitutionnel, alors que cette loi n'a même pas encore été votée. C'est un message négatif transmis à nos forces de l'ordre confrontées aux agresseurs, à la violence des casseurs. Le Président doit clarifier sa position. sa position. Une loi de plus grande fermeté est en voie d'être votée, et nous attendons du Gouvernement, du Président de la République, un soutien sans ambiguïté à nos policiers, à nos gendarmes. Défendre et protéger nos forces de l'ordre ne peut être inconstitutionnel ; l'envisager, c'est déjà les affaiblir ! Le temps de la réflexion et de ce qui a été qualifié de « grand débat » est maintenant derrière nous. Il faut désormais agir, et agir vite. Combien de blessés supplémentaires faudra-t-il avant que ne soit prise la pleine mesure de la situation ? Monsieur le ministre de l'intérieur, voulez-vous continuer à être spectateur des agressions de nos forces de sécurité intérieure, vous qui êtes leur chef ? La proposition de loi du président Retailleau est un texte d'équilibre, doté à la fois d'un volet préventif et d'un volet répressif. Il répond à une attente forte, à une sorte d'appel au secours du terrain pour quiconque écoute et côtoie nos policiers et nos gendarmes. Interdire de manifester à une personne qui a commis des actes violents lors d'une précédente manifestation ou qui présenterait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public relève tout simplement du bon sens. Il s'agit là d'un moyen concret d'écarter les individus les plus à même de commettre des agressions à l'encontre des forces de l'ordre. Lors des précédents mouvements sociaux, la principale difficulté rencontrée par les préfectures et les forces de l'ordre résidait dans l'impossibilité qui leur était opposée de prendre des mesures en amont d'une manifestation. Désormais, il sera possible d'anticiper et de prévenir des atteintes aux personnes et aux biens. Une deuxième mesure consiste à donner davantage de moyens juridiques aux policiers et aux gendarmes. Lorsque cette loi aura été promulguée, le recours aux fouilles de sacs ou de véhicules se trouvera élargi afin d'éviter l'introduction d'armes au sein d'une manifestation. De même, les mesures personnelles d'interdiction de manifester seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées. Ce type de fichage sera immédiatement opérationnel, car la police, la gendarmerie et les douanes disposent de tablettes permettant un accès direct au fichier des personnes recherchées.

puisque ces personnes sont difficilement identifiables hors flagrance. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, les maîtres mots de la proposition de loi de notre collègue Bruno Retailleau sont bon sens et efficacité. C'est la raison pour laquelle je voterai ce texte sans l'ombre d'une hésitation.

Il ressort de nos recherches qu'un certain nombre de manifestations se tiennent sur la voie publique sans que les formalités nécessaires aient été accomplies On se trouve alors dans une zone grise, se situant entre la manifestation légale et l'attroupement, comme l'a dit ma collègue Maryse Carrère lors de la discussion générale, définie par le code pénal en l'absence d'un risque pour l'ordre public. En outre, la marginalisation du fait syndical et l'essor des mobilisations citoyennes annoncées sur les réseaux sociaux rendent ce cadre légal en partie obsolète. Les forces de l'ordre ont déjà adapté leurs pratiques et les renforcent grâce au renseignement en ligne, afin de prévenir les mouvements qui pourraient éventuellement dégénérer. Ces constatations doivent nous inciter à réfléchir à des évolutions législatives plus ambitieuses que celles présentées au travers de cette proposition de loi, qui se concentre uniquement sur les comportements individuels.

afin de rendre le droit au recours des personnes visées par ces interdictions plus effectif, et l'ensemble du dispositif plus opérationnel. Nous sommes conscients que cela pourrait créer, en pratique, une certaine rigidité pour les organisateurs de manifestations,

Néanmoins, le nouveau délai de cinq jours qu'il est proposé d'instituer serait beaucoup plus contraignant pour les organisateurs des manifestations. Il risquerait même de dissuader, encore plus qu'aujourd'hui,

car l'article 2 du texte prévoit qu'une interdiction de manifester devra être prononcée 48 heures avant le début de la manifestation, et non 48 heures après la déclaration.

Fort judicieusement, le Sénat a rejeté, jeudi dernier, la proposition de loi de nos collègues du groupe CRCE qui visait à interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l'ordre.

de se disperser demeurées sans effet. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. Dans les faits, l'autorité annonce sa présence par haut-parleur dans les termes suivants : « obéissance à la loi, dispersez-vous », puis : « première sommation, on va faire usage de la force », et enfin : « dernière sommation, on va faire usage de la force ». Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut-être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge. Or, en plus d'être totalement désuètes, ces modalités de sommation sont très largement inconnues du grand public. S'agissant de mesures réglementaires, je souhaitais interpeller le Gouvernement sur cette procédure, en vue de la rendre plus efficace et plus audible.

? L'amendement n° 10 vise à obliger les organisateurs de manifestations à indiquer, lorsqu'ils déclarent une manifestation, les moyens qu'ils entendent mettre en oeuvre pour informer les manifestants sur les règles relatives aux sommations. Le constat dressé par notre collègue est tout à fait juste : tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le caractère désuet de la procédure de sommations et sur sa méconnaissance par de nombreux citoyens. En revanche, la solution proposée ne me semble pas vraiment appropriée : il appartient aux autorités publiques, plus qu'aux organisateurs, d'améliorer la communication sur les règles de dispersion.

Je crois savoir que le ministère de l'intérieur a engagé une réflexion en vue de revoir la procédure des sommations, ce qui devrait donner satisfaction à notre collègue. Peut-être le ministre pourra-t-il nous en dire davantage à ce sujet

par tout moyen des règles de dispersion des attroupements. Comme je viens de l'indiquer, la commission partage le constat de M. Grand, mais a estimé que le dispositif proposé n'était pas vraiment adapté.

souligner l'importance du volet préventif pour la mise en oeuvre d'une politique de maintien de l'ordre efficace et adaptée. L'article 1 permet de renforcer les actions de prévention des forces de l'ordre, ce qui est une nécessité absolue.

Ces casseurs professionnels ou « cagoules noires » affaiblissent notre République. Ils instrumentalisent le droit de manifester pour agresser, pour saccager, pour piller tout ce qui peut ressembler, à leurs yeux, à un symbole de l'État « capitaliste et policier

sauf à ne pas vouloir considérer que ces groupes anarcho-libertaires, qui déploient leur violence ici et là depuis une vingtaine d'années, ne cherchent qu'une chose : détruire, indépendamment de l'objet de la contestation. preuve non seulement de naïveté ou d'une vision irénique que de croire qu'il n'en est pas ainsi, mais aussi d'un aveuglement idéologique. Tout législateur responsable se doit de pallier les lacunes et les manquements du cadre juridique actuel, en dotant nos forces de l'ordre de nouveaux moyens de droit pour prévenir les violences dans les manifestations. Cet article comporte des mesures de police administrative fortes qui permettront de conférer à l'autorité administrative de nouveaux instruments destinés à prévenir, le plus en amont possible, l'infiltration des manifestations pacifiques par des groupuscules ultraviolents. Il s'agit là de mesures de bon sens, qui permettront d'éviter l'introduction, dans les manifestations, de tout objet susceptible de constituer une arme par destination, dans un objectif de protection des citoyens. Je veux saluer ici nos policiers et nos gendarmes, qui doivent exercer leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles et harassantes. Les mesures introduites par cet article sont attendues tant par nos forces de l'ordre que par nos concitoyens, qui attendent du législateur une action rapide, ciblée et déterminée.

le droit effectif de manifester pacifiquement. Il faut empêcher les casseurs, les extrémistes, les violents de s'introduire systématiquement dans les manifestations pour les détourner. Nous nous sommes inspirés des dispositions qui avaient été

sous contrôle du procureur de la République, bien évidemment, à des fouilles de bagages et de véhicules en vue d'identifier les auteurs d'atteintes à la sécurité des biens ou des personnes ou pour prévenir lesdites atteintes.

et une présomption de détournement d'un objet, mais résulte de la constatation du fait ou d'une preuve tangible d'une intention de détournement. Autrement, je ne vois pas quel objet du quotidien ne pourrait pas constituer une arme par destination

La création d'un nouveau régime de contrôles de police judiciaire spécifique aux manifestations présente un intérêt opérationnel majeur pour les forces de l'ordre, dans la mesure où il offrira beaucoup plus de souplesse pour l'organisation des dispositifs de contrôle. La commission des lois a, en conséquence, décidé de souscrire à la rédaction de l'article 1 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Elle émet un avis défavorable

du parquet, de continuer à donner de nouvelles prérogatives au procureur en matière de garantie des libertés individuelles. Ne pouvant souscrire

Sur réquisitions écrites du procureur de la République et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, il autorise les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationales à les assister pour ces contrôles. À l'origine, la proposition de loi sénatoriale prévoyait également la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent également les assister. Cette possibilité a été supprimée en première lecture par notre commission des lois. Si le maintien de l'ordre ne figure pas dans les missions des policiers municipaux, ceux-ci sont régulièrement appelés en renfort sur des opérations de sécurisation, notamment lors de manifestations des « gilets jaunes » en province, en particulier sur les ronds-points. Troisième force de sécurité, les policiers municipaux voient la mutation de leur profession avancer très lentement, par étapes successives : équipement en caméras-piétons, en munitions, accès aux fichiers, etc.

compte tenu de l'évolution rapide des événements lors des manifestations, ces agents pourraient en effet se trouver impliqués dans des opérations de maintien de l'ordre. Or il s'agit de missions pour lesquelles ils ne sont ni formés ni autorisés à intervenir. Nous ne pouvons donc pas accepter

En tant que législateurs, nous avons le devoir de ne pas céder à l'urgence du moment ou aux passions de l'instant. Légiférer, c'est faire la part des choses ; c'est mettre de la distance entre l'actualité et la loi, au nom de l'intérêt général. Les « unes » de la presse et les journaux télévisés passent et s'enchaînent, le droit reste. Je me permets de vous alerter, car ces lois de circonstance s'accumulent, se superposent et affaiblissent peu à peu notre État de droit. Répondre à la violence par la violence, à la révolte par des lois autoritaires, c'est entrer dans le jeu de ceux qui défient l'État, qui accusent notre démocratie d'hypocrisie et de posture lorsqu'elle affirme être le rempart des droits humains. Une démocratie qui a recours à des lois liberticides pour se défendre prend le risque de perdre son fondement. La manifestation est indissociable de notre histoire. Elle a permis l'avènement de la République en 1789 et celui de la démocratie en 1848. Elle est le terreau des conquêtes sociales, notamment celles de 1936 ou de 1968. Elle a accompagné la libération de Paris, les victoires de la France en Coupe du Monde ou le profond soutien à la liberté de la presse et à la République exprimé en 2015. Le droit de manifester est consacré par l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en fixe d'ailleurs la limite, encadré par la loi de 1935. relève d'une interprétation beaucoup trop zélée de la notion de « trouble à l'ordre public », mentionnée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ne respecte vraisemblablement pas nos droits constitutionnels. En permettant de sanctionner des manifestants sur la base de simples soupçons, il ouvre le règne de l'arbitraire et piétine les libertés publiques. En confiant à une autorité administrative plutôt qu'à une autorité judiciaire la charge de déterminer une sanction, il contrevient à la séparation des pouvoirs et aux garanties apportées par l'ordre judiciaire. En désignant subjectivement qui a le droit de manifester et qui ne l'a pas, cet article est un redoutable outil pour réduire les oppositions politiques au silence. Un tel outil n'a pas sa place dans un régime démocratique. Chers collègues, dans les, Montesquieu disait ironiquement qu'il ne fallait toucher à la loi « que d'une main tremblante ». Il est parfois bon de prendre cette recommandation au pied de la lettre. D'ailleurs, même la main de Jupiter tremble, puisque ce dernier, inquiet, envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour « nettoyer » cette future loi de ses scories autoritaires. Le Parlement se grandirait à éviter le ridicule d'un tel scénario. Alors, oui, défendons la démocratie et la République

appelait à réprimer les participants et organisateurs de rassemblements. Ce texte avait été jugé liberticide et abrogé sous la présidence de

d'obligations de « pointage » à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. La mesure permettrait donc d'empêcher certains individus de se rendre aux manifestations à titre préventif et sans qu'aucune condamnation pénale ait été prononcée à leur encontre. Un tel article porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Comment, en effet, les autorités préfectorales pourraient-elles juger de la culpabilité d'un individu et prononcer des mesures attentatoires à la liberté d'aller et venir au regard de prétendues menaces ? Cette mesure illustre la frénésie sécuritaire qui atteint l'exécutif ; elle n'est qu'un instrument dangereux, qui ouvre la voie à l'arbitraire. L'Assemblée nationale a ensuite complété le dispositif par une énième disposition liberticide : l'extension de la mesure d'interdiction de manifestation pour la personne à l'ensemble du territoire national, pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois. Cet ajout apparaît totalement disproportionné et non justifié par la nécessité de sauvegarder l'ordre public. La nouvelle rédaction de l'article 2 a été décriée par l'opposition, et le président Macron semble lui-même pris de doutes, puisqu'il a préféré saisir le conseil des Sages pour qu'il vérifie la constitutionnalité du dispositif. Mes chers collègues, une telle mesure, particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, n'ayant pas sa place dans notre État de droit, nous espérons sa censure par le Conseil constitutionnel.

Le propre de la loi est de s'adapter à une société qui change, faute de quoi elle devient lettre morte. On entend tout et n'importe quoi : non, avec ce texte, nous n'attentons pas à la liberté de manifester ! Ce droit fondamental est garanti par la Constitution

particulière gravité » par leurs « agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent ». En outre, acte violent ». En outre, le texte précise bien que la mesure doit être proportionnée, le juge administratif opérant un contrôle très strict de cette proportionnalité. ! Il faut être dans le déni de réalité, dans l'aveuglement idéologique ou dans la mauvaise foi la plus totale pour prétendre qu'une telle interdiction pourrait toucher des militants pacifiques en raison de leurs convictions ! Il faut aussi mépriser le juge administratif pour penser que de tels abus de droit ne seraient pas sanctionnés

Je condamne sans ambiguïté toutes les formes de violence. Comme vous, mes chers collègues, j'ai été choqué par les images de policiers agressés, de symboles attaqués, de commerces vandalisés. J'ai vu des gens animés d'un pur désir de destruction, qui doivent être réprimés. Mais on ne peut juger du droit de manifester à la seule aune des débordements qu'il peut entraîner. Les délits et les crimes doivent être punis, mais il n'y a plus de démocratie si le préfet les présume pour interdire l'exercice d'une liberté.

du droit de manifester, pas les actes violents. Il intimide le citoyen, et non le délinquant. Le progressisme affiché n'est sûrement pas tourné vers les libertés publiques. Il est alimenté par un courant hostile aux libertés qui s'appuie sur chaque débordement particulier pour demander la suppression d'une liberté générale.

l'inconstitutionnalité est certaine ... Certes, le rapport du Sénat se montre assez prudent sur ce point, et les représentants du ministère de l'intérieur auditionnés ont écarté tout risque d'inconstitutionnalité, réduisant les modifications apportées à l'Assemblée nationale à de simples mesures opérationnelles. Pourtant, les difficultés constitutionnelles posées par l'article 2 sont remontées jusqu'au Président de la République, qui a choisi de saisir le Conseil constitutionnel pour lever

On voit très bien l'enjeu pour le ministère : éviter, d'une part, la surcharge des services préfectoraux, qui pourraient se retrouver dépassés, et, d'autre part, les stratégies de contournement, consistant à « délocaliser » sa participation à une manifestation. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante en la matière : la limitation de l'exercice d'une liberté fondamentale constitutionnellement garantie doit être « justifiée par la nécessité de sauvegarder l'ordre public » et « proportionnée à cet

ayant justifié l'interdiction administrative et les manifestations interdites. Cet article a, finalement, une vertu : pour la première fois, le Conseil constitutionnel devrait statuer sur la valeur juridique du terme « agissements » sur son caractère suffisamment précis ou non. Mais, en attendant, on se retrouve avec un préfet tout-puissant, qui pourrait très bien- il le fait déjà dans le cadre des interdictions administratives de stade, dont s'inspire l'interdiction administrative de manifester -interdire la participation à toutes les manifestations publiques à des personnes coupables, par exemple, d'avoir dessiné des tags ! Oui, les représentants du ministère ont tenté de nous rassurer, mais il ne faut jamais oublier que si les majorités et les décideurs politiques passent, les mentions juridiques, elles, restent

ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration ou dont il a connaissance. »

des fonctionnaires auraient pu périr dans les flammes du bâtiment public qu'ils défendaient ! Trois suspects ont été arrêtés. La police judiciaire les connaissait. Elle a tout de suite écarté la circonstance aggravante d'agissements commis en bande organisée. Ces trois

de police. Ils sont malheureusement le symptôme d'une déstructuration sociale de notre pays, dont nous devrions aujourd'hui gérer les causes, et pas seulement les effets de façon répressive.

-ont fait l'objet d'une judiciarisation lors des épisodes successifs du mouvement des « gilets jaunes ». Le juge pénal a la possibilité de sanctionner les auteurs de violences d'une interdiction de manifestation ou de déplacement dans le cadre des peines dites « complémentaires », au titre de l'article 131-10 du code pénal. pénal. Je doute que le texte proposé puisse apporter en pratique l'efficacité que vous lui prêtez. Nous sommes devant un texte de circonstance. Le sujet n'est pas comparable à la lutte contre le hooliganisme, et il est difficile de soutenir la constitutionnalité

Il s'interroge sur le fait que des directives des autorités semblent s'inscrire dans la continuité des mesures de l'état d'urgence, comme le relevait M. Leconte à l'instant, que, finalement, le régime d'exception empoisonne progressivement le droit commun et que ce qui se passe en ce moment contribue à poser les bases d'un nouvel ordre juridique fondé sur la suspicion, au sein duquel les droits et libertés fondamentaux connaissent une certaine forme d'affaissement.

fortement contestées plus de dix ans après leur instauration, y compris sur le plan du droit. On se rappelle aussi que certaines et certains ont voulu étendre une mesure analogue aux fraudeurs dans les transports commun ... Il me semble essentiel de revenir sur deux points précis : le dévoiement, déjà prévisible, du dispositif et l'atteinte portée aux droits de la défense. L'Assemblée nationale a supprimé la condition préalable d'une

le caractère d'urgence de ce dernier étant déterminé par le juge. L'Assemblée nationale a cru résoudre le problème en instaurant une présomption d'urgence, mais nous doutons clairement de son applicabilité. Les journées ne font que vingt-quatre heures : avec toute la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas changer cela et instruire dans de bonnes conditions les dossiers. Reste donc la solution d'une procédure

à cet article 2. Ces interrogations ne remettent toutefois pas en cause le bien-fondé de la mesure d'interdiction de manifester. Je rappelle que cette dernière n'aura en aucun cas vocation à concerner des manifestants pacifiques : il s'agit de viser uniquement les personnes les plus dangereuses, qui constituent une menace caractérisée pour l'ordre public. Le préfet de police de Paris m'a par exemple indiqué que de 80 à 100 personnes pourraient être concernées en Île-de-France : nous sommes loin de l'atteinte massive à la liberté de manifester

Seraient visées les personnes qui incitent à des actes violents, en les suscitant ou en les encourageant de façon récurrente. C'est exactement ce qui nous a été dit lors des auditions. Ces agissements répétés pourront être détectés par les caméras de surveillance : on vise précisément les meneurs. Mes propos seront consignés

! Enfin, comme pour toutes les mesures de police administrative, la décision du préfet ne sera pas subjective : son arrêté devra être motivé. Des éléments probants permettant d'établir la menace à l'ordre public devront être apportés. À défaut, la mesure pourra être annulée par le juge administratif.

en tête. Par ailleurs, la menace pour l'ordre public est caractérisée par des agissements antérieurs de l'individu commis à l'occasion de manifestations ayant donné lieu à de graves atteintes aux biens et aux personnes.

Cela donne à entendre que l'action administrative pourrait devenir concurrente de l'action judiciaire contre des casseurs, ce qui ne nous paraît pas pertinent au regard de la gravité des faits concernés. Se pose en conséquence l'épineuse question de l'articulation entre les sanctions administrative et pénale. L'interdiction de manifester peut s'apparenter à une sanction administrative. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire, notamment depuis sa décision du 18 mars 2015 : le cumul de sanctions peut exister à condition qu'il n'y ait pas d'automaticité.

en toute logique, un individu s'étant rendu responsable de violences lors de manifestations dans son jeune âge pourrait théoriquement faire l'objet d'interdictions de manifester plusieurs années plus tard.

fondés sur des notes de renseignement, et des critères « objectifs », tels que l'ouverture d'une procédure devant le juge judiciaire. Cette rédaction se fonde sur le contrôle exercé par le juge administratif en matière d'expulsion des étrangers lorsqu'il évalue la menace grave pour l'ordre public que représente un individu. Enfin, l'amendement vise à établir une sorte de prescription administrative, en prévoyant qu'une personne ne pourra être l'objet d'une interdiction de manifester prononcée sur le fondement d'infractions pénales constatées il y a plus de six mois.

Le seul fait de participer à un attroupement sur la voie publique constitue certes un délit, mais ne paraît pas suffisant pour établir l'existence d'une « menace d'une particulière gravité pour l'ordre public Une personne qui ne se disperse pas après sommations est en situation illégale, mais elle n'est pas pour autant à l'origine de troubles à l'ordre public. En second lieu, retenir la rédaction proposée ne permettrait plus de viser les « meneurs ». Une telle restriction serait fortement dommageable sur le plan opérationnel et limiterait considérablement l'efficacité de la mesure. Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 431-3 du code pénal, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public Si ce flou permet en temps normal une application souple du droit de manifester, il serait en revanche particulièrement problématique qu'une interdiction individuelle de manifester soit prise sur son fondement dès lors qu'il existe une incertitude jusqu'à la tenue effective Dans ce cas, l'interdiction de manifester constituerait une atteinte non seulement au droit de manifester, mais également une atteinte à la liberté d'aller et venir ... Faute d'étude d'impact, nous ne connaissons ni le nombre de manifestations non déclarées en préfecture ne constituant pas un attroupement ni le ratio entre manifestations anticipées par les préfectures

Il est en particulier prévu que le périmètre géographique de l'interdiction de manifester ne pourra comporter ni le lieu de résidence de l'individu ni son lieu de travail. Le présent amendement vise à souligner les difficultés familiales qui pourraient résulter d'interdictions portant sur un périmètre incluant, par exemple, le domicile de parents de l'individu ayant besoin d'être assistés par lui. Dans un sens, la définition du périmètre n'est pas respectueuse du droit de mener une vie familiale normale tel que défini par la Convention européenne des droits de l'homme et interprété par la cour de Strasbourg. L'objet de cet amendement est donc d'y remédier. Quel est donc d'y remédier. Quel est l'avis de la commission ? En première lecture, le Sénat avait exclu du périmètre des interdictions de manifester le domicile ainsi que le lieu de travail de la personne, de manière à se conformer aux exigences constitutionnelles. Par cet amendement, notre collègue souhaite aller plus loin, en excluant également du périmètre le domicile des membres de la famille de la personne faisant l'objet de l'interdiction. Je note que cette précision ne constitue pas ne constitue pas une exigence posée par le Conseil constitutionnel pour garantir le droit à une vie familiale normale. Dans sa décision du 9 juin 2017 qui a censuré les interdictions de séjour de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel n'a ainsi fait référence qu'au domicile

Les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 2 ont été introduites à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement. Elles visent à permettre à l'autorité administrative de prononcer des interdictions personnelles de manifester applicables à tout le territoire national et pour une durée maximale d'un mois. Si l'on comprend la motivation pratique qui sous-tend cette extension du champ de l'interdiction de manifester- il serait en effet relativement facile, pour une personne interdite de manifester dans une ville, de se rendre dans une autre ville pour prendre part à un autre cortège -, une telle mesure suscite d'importantes interrogations. Compte tenu des faibles garanties juridictionnelles prévues dans le texte et de la possibilité, pour le préfet, de prononcer cette interdiction dès lors qu'il « a connaissance » d'une manifestation, même non déclarée, des applications dévoyées pourraient intervenir, qui reviendraient à une forme de déchéance temporaire et partielle de citoyenneté pour certains individus. Néanmoins, l'évolution la plus problématique est l'extension de l'interdiction de manifester dans le temps, qui ne concernait à l'origine qu'une manifestation. Cela rejoint les inquiétudes que nous avons déjà formulées à propos de

Ces deux amendements reviennent sur l'ajout de l'Assemblée nationale visant à autoriser le préfet à prononcer une mesure d'interdiction de manifester valable sur tout le territoire national, pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois. L'extension à tout le territoire de l'interdiction de manifester apparaît utile sur le plan opérationnel. Lorsque plusieurs manifestations sont organisées de manière concomitante sur le territoire, il s'agit en effet d'empêcher une personne interdite de manifester à Paris de se rendre à Lille pour ce faire, par exemple. Il est vrai, en revanche, que l'extension jusqu'à un mois de l'interdiction soulève plus de questions. Néanmoins, des assurances importantes nous ont été apportées sur ce point par les services du ministère de l'intérieur, notamment quant au nombre très réduit de personnes qui pourraient être concernées. C'est pourquoi la commission a décidé d'adopter l'article 2 sans modification.

concerne les mesures limitatives de liberté, qui sont dans le champ de la police administrative, les principes de nécessité et de proportionnalité s'appliquent, même sans texte.

celle-ci n'atteindra que les personnes qui présentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. C'est donc par conviction, en tant que parlementaire, que je me positionne,

pour les actes réglementaires ou de portée collective, il est constant, en droit français, que, pour être revêtue de la force exécutoire, une décision administrative individuelle défavorable doit être notifiée à la personne concernée. En effet, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, « sauf sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ». Dans sa jurisprudence, le juge administratif toutefois fait preuve de souplesse à ce sujet, en considérant que, dans certains cas, une information verbale valait notification. S'agissant de la notification d'une décision pouvant entraîner des conséquences

dès lors qu'il s'agit d'une liberté fondamentale et d'un droit politique, dont l'affaiblissement pourrait s'avérer particulièrement sensible, selon le contexte politique. Quel est l'avis

Il s'agit donc d'assurer l'effectivité, dans la pratique, de la mesure d'interdiction de manifester. Pour cette raison, la

Cet amendement vise ainsi à prévoir qu'une interdiction de manifester ne puisse être prise à l'encontre d'un mineur qu'après un avis préalable du procureur de la République.

il paraît difficile de concilier une procédure d'avis préalable avec les délais très contraints qui s'imposent pour le prononcé de la mesure. l'intervention d'une autorité judiciaire dans le prononcé d'une mesure administrative soulève de nombreuses interrogations quant à sa compatibilité avec le principe de séparation des pouvoirs. On peut en effet se demander dans quelle mesure une autorité judiciaire pourrait intervenir dans un processus de nature administrative, dont le contrôle relève d'un autre ordre de juridiction. Pour l'ensemble de ces raisons, la

Pour la constitution d'un fichier aussi sensible, il semble plutôt curieux que la droite sénatoriale et l'exécutif jugent bon de se passer de l'avis de l'autorité chargée de veiller au respect de la vie privée de nos concitoyens Cet article étant, dans sa rédaction actuelle, particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, nous en demandons évidemment la suppression. Quel

J'observe que les magistrats sont eux-mêmes favorables à ce dispositif, madame Benbassa, car les peines complémentaires d'interdiction de manifester ne figurent actuellement pas au fichier des personnes recherchées. Je précise, enfin, que les modifications opérées par l'Assemblée nationale ne contournent pas l'avis de la CNIL, dès lors qu'il s'agit simplement de compléter un fichier existant. Bien sûr ! Le futur décret modifiant ce